La séance est ouverte. Le compte rendu intégral de la séance du mercredi 24 juillet 2019 a été publié sur le site internet Il n'y a pas d'observation ? ... Le procès-verbal est adopté. J'ai reçu de M. le Premier ministre communication du décret de M. le Président de la République en date du 21 août 2019 portant convocation du Parlement en session extraordinaire à compter du 10 septembre 2019.

Madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, c'est avec une grande émotion que nous avons appris, le 27 août dernier, le décès de notre doyen Philippe Madrelle, qui était sénateur depuis 1980. Souvenez-vous, il s'était exprimé

socialiste et républicain, Patrick Kanner, avec le ministre chargé des relations avec le Parlement et nombre de ses collègues, le 2 septembre dernier, à ses obsèques en l'église Notre-Dame de Bordeaux.

Il fut un militant infatigable de la Gironde, un défenseur du rôle des collectivités territoriales, un socialiste engagé. Souvenons-nous, c'était ici même, le 2 octobre 2017, il nous appelait, dans son discours de doyen, à « prendre en compte la lassitude et les attentes des élus locaux qui animent dans la proximité les cellules de base de la République et de notre démocratie représentative Je souhaite redire ma sympathie et ma compassion à sa famille et à ses proches, ainsi qu'au président et aux membres de son groupe, le groupe socialiste et républicain. Je voulais ouvrir cette session extraordinaire en partageant une pensée pour notre doyen je vous invite à quelques instants de recueillement.

de notre ancien collègue Philippe Leroy, qui fut sénateur de la Moselle de 2001 à 2017, et de celui de notre ancien collègue André Jourdain, qui fut sénateur du Jura de 1989 à 2001. J'informe le Sénat que M. le ministre de l'intérieur a fait connaître que M. Hervé Gillé remplace, en qualité de sénateur de la Gironde, notre regretté collègue Philippe Madrelle. Son mandat a commencé le 28 août 2019. Je lui souhaite, au nom du Sénat tout entier, à l'occasion de l'ouverture de cette session extraordinaire, la bienvenue au Sénat et l'assure

En application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution, ainsi que de la loi organique n° 2010-837 et de la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 prises pour son application, la commission de l'aménagement du territoire a émis, lors de sa réunion du 11 septembre 2019, un avis favorable, par 15 voix pour, à la nomination de Mme Virginie Schwarz aux fonctions de président-directeur général de Météo France. Je rappelle au Sénat que les commissions mixtes paritaires chargées d'élaborer des textes sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l'énergie et au climat et de la proposition de loi relative à la création d'un Centre national de la musique sont parvenues à l'adoption de textes communs.

La délégation est accompagnée par notre collègue Bernard Fournier, président du groupe d'amitié France-Roumanie. Cette visite s'inscrit dans le cadre des échanges interparlementaires que nous entretenons, Sénat français et Sénat roumain, notamment sur la mise en oeuvre du partenariat stratégique franco-roumain, l'actualité européenne et le partenariat oriental. Je le rappelle, le président du Sénat roumain a assuré, avant la France, la présidence des Sénats d'Europe,

État, car c'est la marque de fabrique des Sénats dans nombre de pays. En votre nom à tous, permettez-moi de souhaiter à nos amis roumains un séjour et des échanges fructueux, en formulant le voeu que cette rencontre contribue à renforcer nos liens. Nous leur souhaitons donc la plus cordiale bienvenue au Sénat de la République française

Monsieur le président Gérard Larcher, madame la rapporteure, chère Marta de Cidrac, madame la rapporteure pour avis, chère Anne-Catherine Loisier,

les sénateurs, l'émotion me subjugue, si je puis dire, puisque j'ai peine à parler devant votre assemblée. N'y voyez là aucun signe, si ce n'est du respect et de ma volonté de commencer sur le bon pied Les Grecs nommaient l'art de saisir une occasion au bon moment et de prendre une décision forte. Et c'est ce que j'invoquerai devant vous en cet instant, au moment de vous présenter le projet de loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. C'est en effet le moment d'agir. La planète se dégrade. Nos enfants respirent mal, 200 espèces disparaissent chaque jour et l'artificialisation des terres menace la baisse du réchauffement, tout comme la biodiversité. Les périls climatiques exigent des actes concrets et vous, ici, vous le savez mieux que quiconque. Le temps est venu de prendre

de passer de notre société actuelle, caractérisée par beaucoup d'excès, à une société où chacun peut mieux se déplacer, mieux se loger, mieux se nourrir et vivre dans un environnement plus propre. C'est aussi, car chacun y a droit, C'est, finalement, donner la possibilité à chacun, quelle que soit sa condition sociale, de pouvoir participer à un projet plus grand, celui de la construction d'une société où la prospérité n'est possible que si elle passe aussi par celle de la planète et celle des hommes.

Crise sociale, d'abord, parce que la mondialisation économique, telle que nous l'avons connue depuis les années quatre-vingt-dix, a fait émerger des inégalités sociales croissantes. Nombre de Français se sentent exclus de ses bénéfices et éprouvent un sentiment de perte de contrôle. Crise environnementale, ensuite, parce que nul ne peut désormais ignorer la destruction accélérée de notre biodiversité et la hausse du niveau mondial des émissions de gaz à effet de serre. C'est la raison pour laquelle je suis persuadée qu'une véritable transition écologique ne peut voir le jour dans notre pays que si elle est un instrument de lutte contre la crise sociale. Pendant trop longtemps, nous avons opposé les questions sociales aux questions environnementales. Pire peut-être, nous les avons hiérarchisées, les secondes demeurant l'angle mort des premières, ponctuellement ressuscitées mais jamais au coeur de nos politiques publiques. Mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, sans prétendre épuiser la profondeur de ce vertigineux défi, j'ai la conviction que ce projet de loi anti-gaspillage pour une économie circulaire peut constituer une brique importante pour y répondre dans notre quotidien, sur nos territoires et à l'échelle nationale. C'est la raison pour laquelle je suis persuadée qu'une véritable transition écologique ne peut voir le jour dans notre pays que si elle est un instrument de résorption de la crise sociale. La transition écologique ne sera acceptable par nos concitoyens que si elle est créatrice de richesses économiques, d'emplois, d'amélioration du pouvoir d'achat

après une crise née, notamment, du rejet d'une fiscalité écologique trop lourdement ressentie par les ménages les plus modestes. Nous vivons, dans le même temps, une période de mobilisation sans précédent de la jeunesse en faveur du climat et constatons une sensibilité très forte aux enjeux écologiques Conscients de l'urgence écologique qui les affecte dans leur vie quotidienne- épisodes de chaleur, sécheresse, incendies sans précédent -, les Français exigent, d'une part, des moyens pour agir, chaque jour, à leur échelle, contre le gaspillage des ressources de la planète, et, d'autre part, que les efforts soient équitablement répartis. Ils exigent, en somme, que chacun, citoyen, élu, entreprise, agisse au maximum de ses facultés pour enclencher de nouveaux modes de production, de nouveaux modes de consommation et d'alimentation. Ils nous demandent de construire une société dans laquelle chacun a le « pouvoir de faire », comme le dit Amartya Sen. C'est donc bien le sens et la finalité d'un capitalisme de surconsommation, presque vorace, que les Français interrogent aujourd'hui. Ils nous demandent d'agir pour passer d'une société du tout-jetable à une société économe de ses ressources et respectueuse de l'environnement, à une société du tout-réutilisable. Nous voulons transformer notre système productif pour mettre la préservation des ressources naturelles en son coeur. Cela suppose de supprimer les emballages inutiles, d'encourager le réemploi, de développer la réparation et, en dernier recours, de procéder au recyclage. C'est ce qu'on appelle l'économie circulaire. Elle est l'économie du XXI siècle, celle qui permettra de redonner du sens au capitalisme. L'économie circulaire, c'est aussi une réponse à ceux qui voudraient nous faire croire qu'il n'y a pas d'autre choix qu'entre croissance et décroissance. Je crois qu'il y a une voie médiane et que c'est à nous, collectivement, de la dessiner. Ce projet de loi entend installer un cadre pour transformer notre « pacte productif » et donner aux Français les moyens de consommer autrement. C'est pour répondre à cette attente sans précédent que nous souhaitons désormais nous attaquer à la réduction de toutes les formes de gaspillage, à commencer par celle que constitue la poubelle des Français, car les déchets ne sont pas une rivalité triviale.

Exactement, monsieur le sénateur ! Pourquoi cette passion ? Parce que les déchets disent beaucoup de ce que nous sommes, de qui nous sommes, de notre rapport aux choses et à la nature. Marcel Mauss, un auteur qui m'est cher, disait que c'est « en fouillant un tas d'ordures que l'on peut savoir tout d'une société ». C'est vrai ! Qui peut lui donner tort ? ? Après la révolution hygiéniste du XIXsiècle, qui aura vu l'explosion des déchets des villes, après un XX siècle qui aura été celui de la prolifération des produits à usage unique, nous devons construire un XXI siècle qui sera celui de la consommation sobre, sobre, de la fabrication de produits de qualité faits pour durer des années, en étant réparables, réutilisables et, en fin de vie, recyclables, pour que rien ne se perde plus. plus. Il faut que nos gestes quotidiens sortent de leur mécanique absurde et deviennent des vecteurs de lien avec la nature qui nous entoure plutôt que de saccage de celle-ci. Finalement, il s'agit de remettre du sens dans nos vies quotidiennes. En France, on produit 5 tonnes de déchets par an et par personne, 600 kilos de déchets ménagers, 700 kilos de déchets des entreprises, autant pour le seul secteur du bâtiment, et 2,7 tonnes, plus que la moitié, pour le secteur des travaux publics. Aujourd'hui encore, selon les évaluations les plus conservatrices, 200 millions de bouteilles en plastique sont jetées dans la nature chaque année en France, et seuls 26 % de nos déchets plastiques sont recyclés. Près de trente ans après la dernière grande loi sur les déchets de 1992, on continue encore massivement à envoyer les déchets dans des décharges saturées ou, pire, à les déverser parfois dans la nature, sous forme de dépôts sauvages, voire à les envoyer à l'étranger, dans des pays émergents, comme si ceux-ci pouvaient tolérer longtemps de servir d'exutoires à nos propres excès. Ce projet de loi répond donc à la fois à des enjeux environnementaux, à des enjeux de développement économique et d'emploi et à des enjeux de souveraineté pour la France. C'est cette réconciliation entre le social et l'écologique, entre le développement économique et la protection de l'environnement, que nous demandent les Français. Laissez-moi vous parler des enjeux et des impacts derrière ce projet de loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. évoquant les impacts environnementaux, à la fois en termes de ressources naturelles et de climat. En favorisant le réemploi, la réutilisation, la réparabilité, la longévité des produits, nous voulons réduire la consommation de ressources naturelles et la production de plastique. Nous entrons dans l'ère du post-plastique. C'est la raison pour laquelle les filières REP, pour « responsabilité élargie des producteurs », devront désormais prévoir, dans leur cahier des charges, des objectifs chiffrés de réemploi des matières concernées. De même, les éco-modulations doivent permettre de lutter contre le suremballage, comme l'ont souligné de nombreuses ONG environnementales- je pense à Tara Océan, à Zero Waste et à beaucoup d'autres. Enfin, dans le système de consigne proposé, aucune consigne pour recyclage ne pourra être mise en place sans que les collectivités l'aient décidé. C'est un message que je souhaite affirmer pour avoir entendu les travaux en commission.

pendant la phase de transition et répond à certains défis environnementaux majeurs. En recyclant le plastique, on évite l'importation de pétrole et on réduit les émissions de CO2. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas réduire drastiquement à la source la production de plastique ; j'y reviendrai.

Ce projet de loi est donc au coeur de notre stratégie pour aller vers une société neutre en carbone d'ici à 2050, conformément à l'accord de Paris et aux objectifs qui nous engagent.

pas seulement dans quelques métropoles, mais seraient aussi locaux, territoriaux, non délocalisables. Ce sont aussi des emplois qui couvrent toute la palette de qualifications dans les domaines de l'éco-conception,

Ce sont également de nouvelles opportunités pour l'économie sociale et solidaire, qui représente aujourd'hui 10 % de nos emplois et qui doit prendre plus de place encore. Si ce nouveau modèle nécessite une transformation industrielle profonde, avec de forts besoins d'investissement- 4,5 milliards d'euros pour moderniser et augmenter nos capacités de recyclage sur les cinq prochaines années -, il renforcera les atouts du « made in France », du fabriqué en France, notre indépendance économique, notre indépendance industrielle et, par là même, notre indépendance politique. Enfin, il y a aussi les impacts en termes de souveraineté pour la France. Il faut être cohérent, on ne peut pas, d'un côté, mettre une taxe sur le carbone pour devenir moins dépendant de pays tels que l'Arabie Saoudite et, de l'autre, laisser les ressources nécessaires pour réaliser la transition écologique, par exemple les métaux rares, dans les mains d'autres pays, notamment asiatiques. C'est C'est donc, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, avec autant d'ambition que d'humilité que je suis devant vous aujourd'hui. Ambition, parce qu'il en faut pour relever ce défi, et je sais que vous serez au rendez-vous, vous nous l'avez déjà montré. J'aime à penser que vous et moi, nous sommes comme le Morel de Romain Gary, qui, lui, ne s'est pas désespéré. Humilité aussi, parce que ce combat a commencé il y a longtemps. Je le sais, mes prédécesseurs, de tous les bords politiques, ont déployé des efforts considérables depuis près de trente ans. Je le sais aussi, députés et sénateurs sont engagés depuis de nombreuses années sur ces sujets. sujets. Sur le terrain, au quotidien, maires et élus locaux se battent tous les jours, parfois au péril de leur vie, pour gérer les déchets de leur territoire. J'ai évidemment une pensée à cet instant pour Jean-Mathieu Michel, maire de Signes, dont la mort nous place collectivement face à nos responsabilités. Cela nous rappelle combien les élus locaux, ceux des territoires que vous représentez, qui font la politique de gestion des déchets en France, sont finalement en première ligne sur la transition écologique et solidaire. Ce texte est pour eux. Je m'inscris dans la continuité de cet héritage et je veux rendre hommage à tous ceux qui ont participé à cette grande aventure, celle de la responsabilité élargie des producteurs inscrite dans le droit français dès 1975, celle du « bac jaune celle de l'éducation aux gestes de tri, celle des centres de collecte et de recyclage et des initiatives innovantes qui servent chaque jour l'intérêt général et le bien-vivre sur notre territoire. Oui, nos élus locaux s'attachent à mettre en oeuvre cette politique depuis des années et des années. ces trente années de politique publique, dans la continuité desquelles je m'inscris, ont permis à la France d'être aujourd'hui reconnue pour le travail remarquable qui a été effectué sur ce sujet. Je voudrais, à ce titre, remercier non seulement les élus engagés,

de dîners prolongés, pour discuter et élaborer collectivement ce projet de loi anti-gaspillage. Nous devons aller encore plus loin parce que la donne a changé.

Or, lorsqu'il s'est construit, nous partions presque d'une page blanche. Avoir des objectifs de performance tels que nous les atteignons aujourd'hui était déjà colossal à réaliser. Eh bien, nous l'avons réalisé, avec les élus locaux et les territoires. Nous l'avons fait en France.

l'excellence et ils ont une tolérance zéro pour le gaspillage. Faire ce pas en avant, c'est-à-dire passer de 26 % d'emballages plastiques collectés et recyclés à 90 %, conformément aux exigences de l'Union européenne, cela impose de nouvelles pratiques. Tel est en grande partie l'objet de ce projet de loi.

un gain de 500 millions d'euros par an pour les collectivités. Je parle bien d'un transfert de 500 millions d'euros par an. Entrons dans le détail. Aujourd'hui, la gestion des dépôts sauvages sur les territoires représente pour les collectivités une charge comprise entre 340 et 420 millions d'euros.

Dans des proportions moindres, mais tout de même significatives, la prise en charge des lingettes imbibées coûte aujourd'hui 161 millions d'euros aux collectivités. Pour les jouets, 10 millions d'euros ; pour les produits chimiques non encore couverts par la REP existante sur les déchets diffus spécifiques, 30 millions d'euros ; pour les mégots, 6 millions d'euros ; pour les articles de sport, 14 millions d'euros ; pour les articles de bricolage,

L'objectif de ces nouvelles filières REP est bien de transférer la charge des collectivités vers les industriels et ainsi d'alléger la poubelle de nos contribuables, de nos concitoyens. Ensuite, au-delà de son impact financier, le dispositif mis en place dans le cadre de la REP Bâtiment est profondément en faveur des collectivités. À la suite de la mort du maire de Signes, j'avais annoncé que je réunirais les acteurs de la filière du bâtiment et de la construction, ainsi que des associations d'élus. Chose promise, chose due : une réunion s'est tenue le 5 septembre dernier. Je remercie d'ailleurs certains d'entre vous de leur présence. Cette réunion a été l'occasion de créer un consensus autour de la reprise gratuite des déchets du bâtiment, dès lors que ceux-ci ont été triés au préalable,

Un travail en commun sera mené afin de planifier la localisation de nouveaux points de collecte des déchets pour les professionnels, de manière à densifier le maillage territorial existant. Dans les zones rurales en particulier, il n'y a pas assez de déchetteries : c'est encore un poids qui pèse sur nos élus. activités polluantes, ou TGAP, pour les collectivités qui résorbent leurs décharges sauvages. Ce consensus, atteint dans le cadre d'une concertation responsable, va nous permettre, si vous adoptez cette disposition, de changer durablement la donne pour résoudre une difficulté délaissée depuis des années sur les territoires.

Dès lors que le déchet devient une ressource, dès lors qu'il n'est plus ni brûlé ni enfoui, il constitue une matière première et devient une ressource à exploiter. C'est le cas du plastique, bien sûr : il faut en priorité le réduire à la source- je l'ai dit et nous y travaillerons on estime que le recyclage d'un million de tonnes de plastique permettrait la création de 3 000 emplois industriels. Nous mettons sur le marché 5 millions de tonnes de plastique par an. Le gisement d'emplois dans le recyclage est donc énorme, dès lors qu'on se retrousse les manches. Quelle activité économique peut se prévaloir aujourd'hui d'un tel potentiel d'emplois locaux non délocalisables ? C'est le cas aussi pour la lutte contre l'obsolescence programmée, qui permet de créer de véritables filières de réparation et d'économie de la fonctionnalité sur les territoires. Nous devons encourager la réparabilité

Enfin, ce projet de loi donne aux maires, qui sont confrontés dans leur quotidien à la gestion des déchets, de nouveaux outils pour lutter contre les dépôts sauvages, notamment par le biais du renforcement de leurs pouvoirs de police. Là aussi, nous vous avons écoutés.

programmée, a révélé hier, dans un rapport, que la durée de vie des machines à laver avait diminué de trois ans en moyenne au cours des huit dernières années. Ce n'est pas acceptable.

but est de favoriser le réflexe de réparation chez le consommateur, de mieux structurer les réseaux de réparateurs et, au bout du compte, d'allonger la durée de vie des produits. C'est bon pour la planète, c'est bon pour le pouvoir d'achat et c'est bon pour l'emploi Deuxième axe : donner aux citoyens les moyens d'agir pour la planète en adoptant le bon geste de tri. Il s'agit d'harmoniser au plus vite la couleur des poubelles, comme nous le demandent massivement les Français, et de leur donner une information claire sur le geste de tri.

Ce projet de loi, dans ses articles 7 à 10, transfère, comme je l'ai expliqué, près de 500 millions d'euros aux collectivités. Le Gouvernement a souhaité ce transfert parce qu'il est persuadé

pourquoi il faut donner des moyens aux maires, aux collectivités, et faire en sorte que les industriels du tabac prennent leurs responsabilités et luttent activement contre la pollution causée par les mégots de leurs cigarettes. Il en est de même pour les articles de sport.

c'est la réalité d'une partie de notre système économique. C'est bien à cela que s'attaque le titre III de ce texte, relatif à la lutte contre le gaspillage. L'article 5 prévoit l'interdiction de l'élimination des invendus non alimentaires : c'est une première mondiale ! La France a été pionnière sur le gaspillage alimentaire.

toutes les modifications que vous avez proposées. Loin des clichés, vous avez souhaité, vous aussi, illustrer votre engagement environnemental. Je veux citer, à cet égard, plusieurs des avancées que, de notre point de vue, vous avez apportées à ce projet de loi et sur lesquelles, avec mes services, nous avons travaillé. des dispositions contre la publicité incitant au rebut, le renforcement de la compétence des régions, des précisions relatives aux modalités d'étiquetage, des mesures visant à mieux lutter contre le gaspillage alimentaire,

au premier article de ce texte, d'un amendement porté par le groupe communiste, visant à inscrire dans la loi l'objectif fixé par le Président de la République de 100 % de plastique recyclé. Sur tous ces points, j'applaudis des deux mains.

outre la lutte contre la prolifération du plastique à la source, d'avoir les moyens de faire plus pour lutter contre la pollution plastique. Ainsi, 83 % des Français interrogés souhaitent qu'on leur donne plus de moyens

Mesdames, messieurs les sénateurs, je cherche simplement, en toute humilité, à vous expliquer certains de nos choix. Je sais que certains s'y opposeront,

d'une façon ou d'une autre, à une consigne pour réemploi. Chaque année, en France, malgré les efforts sans relâche et les performances remarquables de certaines collectivités, 200 millions

aux industriels, au travers de leurs éco-organismes, ils n'ont pas toujours honoré leurs engagements vis-à-vis des collectivités. Disons-le ! Je sais que vous le savez. Eh bien, aujourd'hui, ils ont décidé d'avancer de leur côté, sans associer les collectivités. Vous le savez comme moi, car vous l'avez vu sur vos territoires. De grands industriels du secteur agroalimentaire font alliance avec la grande distribution et installent des systèmes de consigne en vase clos, sans en parler aux élus, sans en parler aux collectivités locales. Et vous laissez faire ? Vous avez raison, monsieur le sénateur : nous ne laissons pas faire

trop souvent, en Asie ou ailleurs ? S'ils le savaient, si leurs administrés le savaient, continueraient-ils à faire confiance à certains gros acteurs du secteur ? Je n'en suis pas sûre Des entreprises qui ont pignon sur rue, qui se vantent d'avoir les meilleures performances possible, travaillent-elles en toute transparence, disent-elles aux élus où finissent les déchets ?

Cela fait partie des questions que les Français nous posent et auxquelles nous devons répondre. Il nous faut, mesdames, messieurs les sénateurs, défendre le système public de gestion des déchets. Dans notre projet de loi, nous avions fait le choix d'un principe de consigne large, dont les modalités resteraient à définir avec les parties prenantes concernées.

que soulève ce nouveau système. La version adoptée en commission conduit à laisser le champ totalement libre aux acteurs industriels de la boisson et de la grande distribution. Ils pourraient organiser à leur main, sans concertation, un système de consigne dans lequel les collectivités seraient hors-jeu et n'auraient pas leur mot à dire. Cela est d'autant plus grave que, dans le même temps, de nombreux acteurs industriels se sont déjà organisés pour mettre en place, sans contrainte, ce que le projet initial visait à encadrer.

place, devrait permettre de soutenir et de renforcer les initiatives de consigne pour réemploi. Il n'y a pas d'opposition entre les deux systèmes ; bien au contraire, de nombreuses synergies existent. Aucun système de consigne pour recyclage ne pourra être mis en oeuvre sans qu'il soit adossé, en parallèle, à un objectif de réemploi pour la filière emballage.

On estime même que cela pourrait représenter un gain financier pour les collectivités compris entre 50 et 124 millions d'euros par an selon les hypothèses retenues. Il s'agit là des bouteilles captées par le bac jaune. Troisième principe : les collectivités territoriales doivent être associées à la gouvernance du système de consigne qui sera mis en place. Rien ne pourra être fait sans les collectivités locales.

particulier, pour éviter que ces machines, si elles devaient voir le jour de façon massive, se retrouvent sur les parkings des supermarchés, modèle contre lequel nous nous élevons tous. Soyons cohérents ! Les collectivités doivent également pouvoir, si elles le souhaitent, acquérir des machines et être rémunérées par l'éco-organisme pour le service rendu.

nous assurer que les conditions de mise en oeuvre d'une consigne généralisée, si elle devait voir le jour sur les territoires, répondent bien à une ambition environnementale et à un intérêt économique consigne soit développée de manière complémentaire à notre outil de collecte de tri organisé depuis des années et qui fonctionne très bien, géré qu'il est par les collectivités territoriales. Mesdames, messieurs les sénateurs, j'en arrive au terme de cette longue présentation ... Mais vous n'en avez pas fini avec moi ! Je suis heureuse d'engager avec vous un débat constructif et apaisé. Je veux, pour conclure, vous dire combien ce projet de loi constitue la première brique du nouveau modèle de société que nous devons inventer ensemble : un modèle qui valorise un rapport différent et, oserai-je dire, plus sain, notre environnement et les objets qui peuplent notre quotidien ; une société capable de produire de la richesse à partir de la richesse déjà produite, et non simplement en creusant un peu plus profond encore dans les ressources d'une terre qui exprime presque chaque jour son épuisement une société, aussi, qui crée des emplois pour tous, une société qui a du sens, grâce à une nouvelle économie, une société progressivement libérée du plastique, une société écologique qui partage les responsabilités pour ne pas faire peser sur quelques-uns seulement la charge des excès de tous les autres. Nous aurons, bien sûr, des discussions sur des détails ; nous aurons parfois, je le sais, des désaccords. Mais il nous appartient ici, au-delà des habitudes et, parfois, des rentes, de ne pas perdre de vue cette grande ambition, parce que, là encore, comme disait Romain Gary, « l'inaccessible, on le fabrique soi-même

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, le projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, dont nous commençons aujourd'hui l'examen, doit porter un message clair. En tant que rapporteure de ce texte, je nous appelle collectivement à être au rendez-vous et à ne pas nous tromper de message. L'épuisement de nos ressources naturelles, la dégradation toujours plus rapide de nos écosystèmes, le réchauffement climatique, ou ou encore l'accumulation de déchets plastiques dans nos océans ne nous laissent pas le choix : nous devons aller plus loin dans notre façon de gérer nos déchets, mais nous devons surtout agir sur la prévention. Comment produire moins de déchets ? Voilà la vraie question. Voilà ce qui nous fera sortir vraiment de l'ère du tout-jetable, ce que nous appelons tous de nos voeux, madame la secrétaire Votre texte a été déposé sur le bureau du Sénat le 10 juillet dernier et envoyé à notre commission au fond. Je ne reviens pas sur les mesures qu'il comporte, puisque vous les avez bien présentées à l'instant. Je ne vous cache pas, en revanche, que nous avons été nombreux, au sein de notre commission, à être déçus par son manque d'ampleur. Le Gouvernement auquel vous appartenez a placé haut les ambitions et les espoirs portés par ce texte. Le Premier ministre a lui-même souhaité en faire le premier acte de « l'accélération écologique » du quinquennat. En réalité, il semble que ce projet de loi présente une double faiblesse. Premièrement, les mesures qu'il comporte sont pour une grande partie techniques et viennent prolonger des dispositifs déjà existants. C'est vrai ! Deuxièmement, il n'assume pas d'orientations claires.

comme l'interdiction de la destruction des invendus ou encore la création de nouvelles filières REP. En effet, vous avez vous-même fait de la consigne, madame la secrétaire d'État, le « symbole » de votre texte, alors que le dispositif de consigne pour recyclage sur les bouteilles en plastique envisagé par le Gouvernement nous paraît au contraire, au mieux, anecdotique, au pire, à rebours des véritables défis environnementaux du XXI siècle. Très bien ! Ni concertée ni évaluée, Ni concertée ni évaluée, cette mesure revient pour nous en réalité à donner une prime à la production de plastique et à sanctuariser, dans le même temps, la consommation de produits en plastique à usage unique. Le cas de l'Allemagne, souvent pris en exemple comme pays ayant atteint l'objectif européen des 90 % de recyclage grâce à la consigne, montre que la mise en place de cet outil a coïncidé avec une augmentation de la consommation des emballages et des contenants en plastique à usage unique. Ce n'est pas un hasard si les associations de protection de l'environnement se sont publiquement positionnées contre ce projet de consigne. Comment vouloir, madame la secrétaire d'État, sortir de la société du tout-jetable avec un projet de loi centré sur le recyclage des bouteilles en plastique ? Comment ne pas y voir également un recul dans la prise de conscience écologique, puisque se retrouve « monétarisé » un geste essentiel, aujourd'hui gratuit. Le consommateur vertueux, qui paye aujourd'hui un euro sa bouteille en plastique et la jette dans le bac jaune, devra demain la payer 15 centimes de plus, voire peut-être prendre sa voiture pour la rapporter dans un supermarché. Où est la vertu écologique ? En outre, la mise en place de cette consigne créerait de manière sous-optimale deux systèmes de collecte concurrents : le premier sur l'ensemble des emballages plastiques, financé par les contribuables la collecte séparée, le second sur les seules bouteilles plastiques, financé par les consommateurs la consigne. Cette dernière impliquerait une infrastructure lourde, coûteuse et ultraspécialisée de collecte, alors que le service public de gestion des déchets est déjà déployé dans la France entière et que sa polyvalence lui permet de traiter de plus en plus d'emballages différents, ce que ne permettront pas les machines de déconsignation des bouteilles. D'un point de vue économique, la consigne entraînerait une ponction sur les consommateurs de 150 à 200 millions d'euros et aurait un impact financier négatif sur les collectivités territoriales gestionnaires de déchets, qui pourrait atteindre 150 millions d'euros, avec, en outre, une prime à la sous-performance, puisque ce sont les collectivités les plus performantes en matière de collecte sélective qui seraient mécaniquement les plus pénalisées. la secrétaire d'État, j'ai eu de nombreux échanges avec les associations d'élus locaux comme de consommateurs : elles ont publiquement exprimé leur soutien aux travaux de la commission J'en viens à l'important travail réalisé par notre commission. Je salue d'ailleurs l'ensemble de ses membres, issus de l'ensemble des groupes politiques, qui y ont largement contribué, ainsi qu'Anne-Catherine Loisier, rapporteure de la commission des affaires économiques, saisie pour avis 164 amendements ont été adoptés et le projet de loi comporte désormais 36 articles. Premier axe de travail, la commission a élargi le texte à la lutte contre l'ensemble des déchets plastiques, les seules bouteilles en plastique représentant moins de 10 % de ces déchets. Elle a introduit des mesures importantes visant à lutter contre le suremballage : la mise en place par les pouvoirs publics d'une trajectoire pluriannuelle de réduction de la mise sur le marché d'emballages l'obligation pour les entreprises les plus consommatrices d'emballages de réaliser des plans quinquennaux de prévention et d'éco-conception ; un malus financier pour les entreprises qui suremballent. Notre commission a également souhaité renforcer la collecte séparée « hors foyer » l'affectation d'une partie des contributions financières versées par les producteurs. Elle a interdit la distribution gratuite des bouteilles d'eau plate en plastique dans les établissements recevant du public et dans les locaux à usage professionnel. Au regard de l'impact environnemental et sanitaire considérable de certains produits sur les milieux aquatiques, la commission a souhaité responsabiliser les producteurs de ces produits en les incitant à améliorer la conception de leurs produits ou à financer des opérations de nettoyage des milieux et de traitement de la pollution des eaux. la commission a souhaité renforcer l'information du consommateur, afin de l'inciter à être toujours plus éco-responsable. C'est dans cette perspective qu'elle a souhaité pénaliser l'apposition d'informations environnementales entretenant des confusions dans l'esprit du consommateur, comme le « point vert », qu'elle a facilité l'accès aux informations environnementales figurant sur les produits leur dématérialisation, qu'elle a mis fin aux pratiques publicitaires visant à encourager la mise au rebut de produits encore en état de marche et qu'elle a renforcé la lutte contre le gaspillage alimentaire. Troisième axe de travail, la commission a décidé de mettre l'accent sur la promotion du réemploi.

Elle a favorisé le recours à la filière du réemploi dans le cadre de la commande publique. La commission a également créé un fonds de réparation permettant de prendre en charge une partie des coûts de réparation des produits par des réparateurs labellisés, identifiables par un annuaire en ligne. Elle a enfin fixé des objectifs de réparation au sein des cahiers des charges des éco-organismes. Sur la question des déchets du bâtiment, qui représentent près de 15 % des déchets produits en France, la commission a choisi de conserver le principe de la création d'une nouvelle REP assorti d'une faculté pour les professionnels concernés d'y déroger par un système équivalent, permettant d'assurer la reprise gratuite des déchets. En revanche, elle a souhaité encadrer ce système par des obligations de maillage territorial des points de reprise, d'accessibilité de ces points et de traçabilité des déchets. En outre, elle a prévu que les professionnels du bâtiment devront remettre au maître d'ouvrage un certificat de traitement des déchets induits par les travaux que ce dernier fait réaliser. commission a également souhaité renforcer les moyens permettant de lutter contre les dépôts sauvages, notamment un renforcement des pouvoirs de police des maires, un renforcement de la REP des véhicules hors d'usage ou encore un financement du nettoyage de ces dépôts sauvages par les éco-contributions acquittées par les producteurs. La commission a également étendu la nouvelle filière à responsabilité élargie du producteur prévue pour les lingettes pré-imbibées à l'ensemble des textiles sanitaires. Elle a aussi renforcé la prévention et la gestion des déchets outre-mer une majoration du barème national. en quelques mots, mes chers collègues, les travaux de notre commission. Madame la secrétaire d'État, nous nous retrouvons, je crois, sur les objectifs que nous souhaitons nous fixer pour aller vers une économie circulaire. Les moyens que nous proposons de mettre en oeuvre pour y arriver diffèrent parfois. En tout état de cause, je ne doute pas que nos débats nous permettront d'enrichir encore ce texte important. J'espère que nous nous rejoindrons sur de nombreux points dans l'intérêt collectif,

L'économie circulaire, longtemps abordée par petites touches isolées dans des textes relatifs à l'environnement, à l'agriculture ou à l'énergie, se voit enfin consacrer l'attention qu'elle mérite et je salue votre initiative en ce sens, madame la secrétaire d'État. Plusieurs mesures de ce projet de loi vont dans le bon sens. C'est le cas de l'amélioration de l'information du consommateur, de l'éco-modulation, de l'interdiction de l'élimination des invendus, de l'indice de réparabilité ou de l'affichage de la disponibilité des pièces détachées. Je ne m'y attarderai pas plus longuement et me concentrerai sur trois points. Tout d'abord, l'absence d'études d'impact sérieuses et de perspectives clairement définies fragilise ce projet de loi. Ce texte constitue malheureusement un nouvel exemple du peu de considération pour les études d'impact.

d'État, l'étude d'impact ne doit pas être une formalité administrative. C'est le fondement de l'action, l'assise du projet de loi, une exigence constitutionnelle, un devoir vis-à-vis de nos concitoyens, mais aussi et surtout un enjeu de crédibilité et de compréhension des gouvernants. De même, le législateur ne peut se prononcer sur des textes aux contours incertains, sur des ordonnances pléthoriques mettant en oeuvre des dispositifs dont nous ne connaissons pas la teneur. Les conséquences sont lourdes pour une entreprise qui doit, par exemple, incorporer 50 % de matière recyclée dans un produit ou pour une filière entière devant se conformer aux exigences de la responsabilité élargie du producteur en seulement quelques mois. Dans le cas de la consigne, les approximations du projet de loi sont patentes et nous n'avons toujours pas à ce jour de réponses quant aux modalités mêmes de sa mise en oeuvre sur des sujets fondamentaux comme celui du financement du service public ou encore de la TVA sur la consigne. ce texte attendu s'empare d'un sujet majeur, la gestion des déchets. Mais de nombreux reproches portent sur l'absence de mesures de prévention, sur la question des usages et de la responsabilité même du citoyen. Autant de sujets qui Enfin, sur ce sujet comme sur bien d'autres, la France se veut vertueuse et exemplaire, ce à quoi nous souscrivons tous. Pour autant, nous connaissons à présent les effets ravageurs sur notre économie des surtranspositions de directives européennes. Tout à fait ! Le juste équilibre est donc à rechercher, en prenant garde aux excès franco-français Le mieux étant l'ennemi du bien, nous avons tout intérêt à accompagner nos entreprises dans des efforts d'adaptation plutôt qu'à les fragiliser sans tenir compte des réalités des marchés européens et mondiaux désormais ouverts. Imposer des obligations excessives à nos producteurs et, dans le même temps, autoriser l'importation de produits moins exigeants, nous le savons, n'est pas tenable. Face aux obligations nouvelles, le Gouvernement devra aussi s'engager à dédier de nouveaux moyens de contrôle et de respect des normes. En ce sens, la commission des affaires économiques a été attentive aux équilibres entre enjeux environnementaux, faisabilité économique et technique pour les producteurs, protection des consommateurs, pérennité et financement des missions assurées par les collectivités. Nombre de nos entreprises sont citoyennes et responsables. Elles n'ont pas attendu ce texte pour faire évoluer leurs modes de production au regard des objectifs nationaux et européens, parce que, très prosaïquement, l'environnement est aujourd'hui aussi un argument commercial. Bravo ! Soyons donc pragmatiques et ne détruisons pas ce qui fonctionne bien, privilégions l'obligation de résultat. Ainsi, l'éco-organisme n'est pas l'alpha et l'oméga de la gestion des déchets. Certains secteurs ont développé des alternatives efficaces et exemplaires, comme la filière de l'agrofourniture, qui affiche des taux de collecte impressionnants, bien au-delà des exigences européennes. Bravo ! Je défendrai donc un amendement validant ces initiatives « troisième voie » au sein de la REP. Les filières qui le souhaiteraient pourront ainsi mettre en place un système alternatif, sous conditions, bien évidemment, de l'atteinte des objectifs et d'un contrôle renforcé

une consigne pour recyclage aura des effets préjudiciables et déséquilibrera tout le système collectif existant. Un certain nombre d'incertitudes demeurent, relatives au bilan environnemental, au pouvoir d'achat du consommateur, à l'attractivité du petit commerce ou encore à la participation au financement global du service

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, dans le cadre de sa mission de veille sur les surtranspositions- désormais inscrite dans notre règlement -, la commission des affaires européennes a formulé plusieurs observations sur les dispositions du projet de loi qui transposent les directives adoptées au mois dans le cadre du paquet Économie circulaire, complété, au mois de juin dernier, par la directive concernant certains produits en plastique. Ce paquet fixe des objectifs chiffrés de recyclage, aux horizons 2025 et 2030. Il s'agit d'objectifs globaux, déclinés par matières- avec un accent particulier sur le plastique -et par secteurs. Il précise et renforce le cadre européen, notamment en matière de collecte séparée des déchets municipaux et des biodéchets, ou encore de responsabilité élargie des producteurs. Fondées sur le principe du pollueur-payeur, trois nouvelles filières de traitement devront en outre être mises en place. Certaines prescriptions européennes sont impératives, comme l'interdiction de mise sur le marché de produits à base de plastique oxodégradable ou la mise en place de systèmes de reprise, de collecte et de valorisation des emballages et déchets d'emballage en vue de leur réemploi. Le projet de loi les reprend strictement. La commission des affaires européennes a toutefois constaté que ce texte anticipe la date d'application d'une obligation en matière de traitement des emballages de la restauration rapide. Le texte prévoit en outre des mesures d'application

En revanche, il va au-delà des obligations européennes dans plusieurs domaines, en particulier en matière de garanties financières requises pour l'agrément des éco-organismes, de prise en compte des coûts de nettoyage et de certains coûts de prévention des déchets dans le calcul de l'éco-contribution ou encore en ce qui concerne le champ de l'obligation de reprise des produits usagés. Les directives renvoient en outre aux États membres le soin de prendre des « mesures appropriées », qu'elles encadrent, pour atteindre les objectifs qu'elles fixent. Elles formulent des préconisations ou des suggestions pour faciliter l'atteinte de ces objectifs. Ces mesures ne sont pas imposées par le droit européen, mais s'inscrivent dans la logique d'atteinte des objectifs européens de réduction de la production de déchets et de lutte contre le gaspillage. Le projet de loi en reprend plusieurs : l'information du consommateur sur les qualités environnementales des produits, leur réparabilité et la disponibilité des pièces détachées, l'interdiction de la destruction de certains invendus non alimentaires ou encore le renforcement des conditions d'établissement du diagnostic sur le caractère réutilisable des produits et déchets dans le secteur du BTP. Pour favoriser le recyclage, ce texte introduit en outre un taux minimum d'incorporation de matières recyclées dans certains produits. Il prévoit la création de cinq nouvelles filières de traitement purement nationales et introduit la faculté de mettre en place des systèmes de consigne pour les bouteilles en plastique contenant des boissons. La commission des affaires européennes rappelle que ces surtranspositions doivent être justifiées et examinées, tout comme doivent l'être leurs conséquences sur la compétitivité des opérateurs économiques- producteurs et distributeurs -établis en France, les collectivités territoriales et les consommateurs. Elles génèrent en effet un accroissement des coûts de production et de distribution des produits ainsi que des coûts de collecte des ordures ménagères. Elles imposent de modifier certaines filières de production et risquent dès lors de conduire à une augmentation du prix des produits et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. votre audition, je vous ai rappelé qu'il était impératif que toutes ces conséquences soient évaluées au regard des objectifs européens et nationaux fixés et que ces mesures n'introduisent pas de distorsions de compétitivité de nature à pénaliser les opérateurs français par rapport à leurs concurrents européens. À cet égard, je crains qu'il ne suffise pas de considérer, comme vous me l'avez indiqué, que « les filières REP visent tous les producteurs, qu'ils soient établis en France ou à l'étranger ». Encore faut-il procéder à une analyse détaillée et mesurer l'impact des mesures hors filières, en particulier les coûts non supportés par les producteurs ou distributeurs étrangers pour les produits qu'ils ne proposent pas sur le marché français. ailleurs, je ne pense pas non plus que le renvoi à des ordonnances, dont le contenu n'est pas précisément documenté en l'état, soit une réponse au risque de surtransposition. En conclusion, le bien-fondé des objectifs n'est pas contestable tout est dans la mise en oeuvre. C'est bien sous cet angle que la commission des affaires européennes a souhaité attirer l'attention sur les surtranspositions qu'elle a identifiées dans ses observations. Très bien ! La parole est

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, dans le monde, 10 tonnes de plastique sont produites chaque seconde, consommant 8 % de la production mondiale de pétrole. 9 milliards de tonnes de plastique ont été accumulées depuis 1950. En France, 800 millions de tonnes de déchets sont produites chaque année, soit 25 kilos par seconde. Le plastique représente quant à lui 3 millions de tonnes jetées en France. Ce matériau, qui met des siècles à disparaître, doit donc faire l'objet d'une politique publique ambitieuse et ce projet de loi doit y participer. Bien conscients de ce constat et de la part active qu'ils y prennent en tant que citoyens, les Français ont massivement évoqué le sujet des déchets lors de leur participation au grand débat. Comme le souligne l'exposé des motifs de ce projet de loi, ils exigent des moyens pour agir à leur échelle. Mais ils appellent également à un changement de paradigme de grande ampleur, un changement à la hauteur de l'enjeu. Rappelons qu'un continent de plastique de 1,6 million de kilomètres carrés flotte actuellement dans l'océan Pacifique. Pour réduire la pollution et notre empreinte écologique, la première des solutions est de limiter à la source la production de déchets et le gaspillage. Le groupe du RDSE se joint évidemment à l'ambition du Gouvernement en la matière et salue certaines avancées obtenues en commission la semaine dernière. En ce qui concerne les invendus des produits non alimentaires, il apparaît essentiel d'introduire des sanctions, mais aussi de réaffirmer la hiérarchie des modes de traitement, le recyclage ne devant intervenir qu'en cas d'impossibilité de réemploi ou de réutilisation. Nous devons à tout prix éviter que des produits neufs se retrouvent dans le circuit des déchets. C'est pourquoi nous défendrons un amendement afin d'interdire explicitement tout acte visant à rendre les invendus impropres au réemploi. Complétant ces mesures de lutte contre le gaspillage, notre groupe présentera des amendements visant à limiter la production de plastique, d'abord, en interdisant la mise sur le marché de certaines bouteilles en plastique, ensuite, en interdisant l'utilisation d'emballages à usage unique pour les repas pris sur place dans les établissements de restauration, enfin, en interdisant la mise à disposition de bouteilles d'eau, dosettes et emballages en plastique dans les administrations, considérant que celles-ci doivent être exemplaires en la matière. L'information du consommateur permettra par ailleurs d'orienter ses choix vers des produits écologiquement plus vertueux. Les apports du texte semblent aller dans ce sens. S'agissant du geste du tri, l'accompagnement doit se faire de manière plus lisible et transparente, car les diverses signalétiques perturbent le consommateur. Nous soutenons donc les avancées de ce texte et en appelons à la bonne volonté des producteurs pour enfin faire apparaître ces informations de manière claire et lisible. Nous saluons bien sûr la création de nouvelles filières à responsabilité élargie du producteur, qui transfèrent la responsabilité de la gestion des déchets au producteur et incitent à l'éco-conception. L'établissement d'un cadre commun à toutes les filières permettra par ailleurs d'améliorer leurs performances environnementales. Parmi les nouvelles filières, celle du BTP attire particulièrement l'attention, et pour cause ! Le secteur du bâtiment produit environ 45 millions de tonnes de déchets chaque année, dont la moitié seulement est valorisée. Une large part fait d'ailleurs l'objet de dépôts sauvages, dont le coût de collecte pèse sur les finances publiques, puisqu'il est estimé à 340 millions d'euros par an. Les précisions de la commission en matière de maillage territorial et d'horaires d'ouverture des points de collecte permettront, je l'espère, d'assurer le tri le plus large de ces déchets. Le groupe du RDSE se réjouit d'ailleurs des mesures introduites directement dans le texte concernant la lutte contre les dépôts sauvages. Très seuls face à ces incivilités qui menacent l'environnement et la sécurité des citoyens, les maires verront, je crois, ce soutien d'un bon oeil. Les mesures relatives à l'économie circulaire, qui répondent au paquet européen adopté au mois de mai 2018 et qui reprennent une partie des mesures de la feuille de route pour l'économie circulaire établie à la même période, offrent des perspectives intéressantes en matière de réemploi. J'en ai déjà évoqué quelques-unes. J'y ajouterai celles qui sont relatives à la réparabilité des biens et à la disponibilité des pièces détachées, qui devraient permettre de faire baisser le nombre de déchets et, par la même occasion, les besoins en matières premières. En allongeant la durée d'utilisation d'un bien, on augmente aussi le pouvoir d'achat des ménages et on développe les emplois non délocalisables. Considérant que l'économie circulaire doit être davantage soutenue, nous avons déposé des amendements visant à augmenter encore la part de biens issus du réemploi dans la commande publique et à inciter les collectivités et les administrations publiques à signer des conventions avec des structures de l'économie sociale et solidaire pour favoriser le don de matériels. Ces propositions seront complétées par la mise à disposition, par l'État, d'outils d'analyse du coût du cycle de vie des biens. Ce coût global prend davantage en compte l'impact environnemental, mais aussi la fin de vie du bien et son potentiel de réutilisation. le simple prix d'achat ne peut plus être notre seule base de calcul. L'économie circulaire appelle à un profond changement dans les méthodes de production et de consommation. Pour que ce changement s'opère, nous sommes convaincus que l'action publique doit être aux avant-postes. Je terminerai par le sujet qui a concentré une bonne partie des débats et suscité un nombre impressionnant de sollicitations extérieures. Si nous devions soutenir une consigne, c'est bien sûr celle pour réemploi. Néanmoins, nous nous étonnons de voir cette pratique encadrée, tandis que la consigne pour recyclage est entièrement laissée aux mains des industriels. Nous sommes tous d'accord pour affirmer que la consommation de plastique ne doit pas être encouragée. Les craintes des collectivités doivent aussi être entendues, notamment les plus vertueuses d'entre elles, qui maillent le territoire et pourraient pourtant être les plus pénalisées, d'autant que la rédaction initiale de la mesure ne donnait aucune garantie sur l'encadrement du dispositif. Néanmoins, force est de constater que le système actuel n'atteint pas ses objectifs et, surtout, que des initiatives se multiplient. Veillons donc à ne pas donner toute liberté aux industriels de l'appliquer sans contreparties satisfaisantes. Nous espérons avoir un débat équilibré sur ce sujet, afin d'encadrer les pratiques et de ne pas pénaliser les collectivités, qui, depuis longtemps, consentent des efforts importants en la matière. La parole

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, le groupe Les Indépendants se réjouit que le Sénat soit la première chambre à examiner ce projet de loi contre le gaspillage. Le gaspillage et les déchets qui en sont issus sont en effet une source majeure de pollution, notamment pour nos territoires. Oui, ce sont bien nos territoires qui sont en première ligne dans la gestion des déchets, y compris dans la lutte contre les dépôts sauvages. Comme beaucoup d'entre vous, j'ai une pensée pour Jean-Mathieu Michel, qui y a laissé sa vie.

tous -sont mobilisés pour la préservation de notre environnement, l'environnement de nos concitoyens. Des progrès considérables ont été accomplis ces dernières années. Les élus font beaucoup, mais ils ne peuvent pas tout faire. Nous estimons qu'il n'est pas du tout juste que les collectivités aient à gérer et à supporter le coût des déchets que certains abandonnent sans aucun respect. Nous apprécions ainsi que la gestion des dépôts sauvages échoie désormais aux entreprises soumises à la REP, à la responsabilité élargie du producteur. Plus globalement, il est juste que tous les acteurs concernés soient impliqués et contribuent à l'effort : État, industriels, consommateurs ... Ainsi, nous nous félicitons que de nouvelles filières soient soumises à ce régime, particulièrement celles des produits du tabac, au regard du nombre invraisemblable de mégots qui polluent nos terres

J'ai d'ailleurs déposé un amendement visant à soumettre l'ensemble des producteurs à ce régime, quelle que soit leur filière. Il me semble plus juste que, le plus vite possible, tous y soient soumis. Il me semble également que l'efficacité de ce dispositif s'en trouverait renforcée. Si ce régime nous semble avantageux, il n'est pas parfait pour autant. La gouvernance des éco-organismes n'est pas optimale. Dans le passé, des aventures malheureuses se sont produites. De trop nombreux témoignages font encore état de pratiques discriminatoires. Il faut s'assurer que l'éco-organisme ne puisse pas être le moyen pour certains industriels de contourner la nécessaire libre concurrence. les dispositions du projet de loi sur ce sujet vont dans le bon sens, mais nous pensons qu'elles ne vont pas assez loin. Nous tenterons d'enrichir au mieux le texte sur ce point. Une régulation des éco-organismes serait nécessaire. La création d'une autorité administrative indépendante ou d'un organisme adéquat chargé de veiller au respect des obligations de chacun pourrait être une solution adaptée. L'article 40 de la Constitution rend impossible la proposition d'une mesure de ce type, mais il serait

Ainsi, nous saluons les dispositions du texte portant sur l'information du consommateur. Elles vont vers plus de transparence et plus de responsabilité de chacun. Plus encore, nous sommes convaincus que l'information est toujours

La commission a fait le choix de limiter une éventuelle consigne au réemploi et de ne pas permettre la mise en place d'une consigne pour le recyclage- je salue à cet égard l'important travail accompli par Mme de Cidrac et par Mme Loisier

Nous avons dû travailler dans des délais trop courts, à la sortie de l'été. Fallait-il fermer la porte au recyclage ? Pour le savoir, et pour réfléchir aux meilleurs moyens de lutter contre la pollution,

Madame la ministre, le Gouvernement semble poursuivre sans relâche un objectif : baisser le pouvoir d'achat des retraités ! Il y a eu la hausse de la CSG il y a eu la sous-indexation des retraites ; et maintenant ce sont les déductions fiscales accordées aux personnes âgées de plus de 70 ans employant une aide à domicile qui sont dans le collimateur. Décidément, la personne âgée est bien malmenée par ce gouvernement ! Priver les personnes âgées des moyens qui leur permettent d'être accompagnées dans leur vie quotidienne serait une double erreur, mais sans doute allez-vous nous confirmer que vous renoncez d'abord parce que le vieillissement de la population appelle des réponses multiples. Le rapport Libault, comme le mien du reste, a démontré, s'il en était besoin, que le maintien à domicile reste une priorité absolue pour le bien-être des personnes âgées et pour l'équilibre des finances publiques. Ce serait une faute ensuite parce que faire des retraités les nouveaux boucs émissaires n'est pas digne ! Les personnes âgées méritent notre respect. Vous ne pouvez pas les considérer comme une variable d'ajustement budgétaire.

qu'il n'était pas favorable à l'éventuelle suppression de niches fiscales en faveur des emplois à domicile. On ne peut qu'être d'accord. J'espère, madame la ministre, que cet épisode de va-et-vient, peu glorieux pour le Gouvernement, vous éclairera sur le sens que vous devez donner à la réforme des retraites pas toucher au pouvoir d'achat des retraités. Nous espérons tous, madame la ministre, ... Il faut conclure ! ... que cette volte-face sera l'occasion pour le Gouvernement de renforcer tout ce qui contribue au maintien des personnes âgées à leur domicile. Pouvez-vous nous dire où en est le Gouvernement sur ces sujets ?

Madame la ministre, en tant que médecin, vous mesurez à quel point les personnels soignants sont engagés dans l'exercice de leur métier. Cet engagement profond s'apparente le plus souvent à de l'abnégation. Nous le saluons bien bas. personnels sont à bout : impossibilité de prendre leurs jours de repos, heures supplémentaires pas toujours payées, sous-effectifs, dépressions, burn-out, risques d'erreurs médicales accrus. Le triste accident survenu aux urgences psychiatriques de Niort le dimanche 15 septembre, en raison de l'absence d'un service de sécurité de jour, en est une terrible illustration. La crise des urgences n'est certes pas nouvelle. Le nombre de passages annuels a doublé en vingt ans et triplé depuis 1988. 1988. La situation, qui s'est aggravée d'année en année, est aujourd'hui critique : manque de lits aux urgences et dans les services appropriés, effectifs insuffisants, revalorisation salariale inexistante. Le pacte de refondation des urgences que vous avez présenté il y a quinze jours ouvre certes des pistes intéressantes, mais force est de constater qu'il ne répond pas à l'ensemble des besoins des personnels de santé. La grève se poursuit. Envisagez-vous des mesures complémentaires et nouvelles afin de débloquer cette situation

Je ne reviendrai pas sur les causes de la saturation des services d'urgence. Le constat est connu et partagé par tous ici. Je vous parlerai de l'avenir et des solutions que nous mettons

Outre la création d'un nouvel office spécial, l'Ofast, vous avez annoncé la reconduction du plan d'action interministériel lancé en mars dernier pour renforcer la lutte contre le trafic de stupéfiants en provenance de Guyane. Pour rappel, ce trafic représenterait, selon l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies, près de 30 % du marché français, évalué entre 25 et 30 tonnes. Dans le même temps, en Guyane, les réseaux sociaux, puis la presse, ont révélé que, le 5 août dernier, un colis contenant 8 kilos de cocaïne avait été retrouvé « par hasard » sur la coque du cargo, navire essentiellement dédié au transport d'éléments de la fusée Ariane entre Kourou et l'Hexagone. Je dis bien : « par hasard », puisque le colis aimanté à la coque du cargo se serait détaché seul, attirant ainsi l'attention du personnel du port de Pariacabo, qui a donné l'alerte aux autorités. Je ne suis pas de ceux qui s'émerveillent de l'ingéniosité des trafiquants. Je suis plutôt de ceux qui s'inquiètent qu'une telle information soit découverte plus d'un mois après les faits. Je suis de ceux qui sont ahuris par le fait qu'un cargo puisse quitter un port aussi surveillé que celui de Kourou, principalement utilisé pour les besoins du Centre spatial guyanais, avec à son bord du matériel spatial et de la cocaïne Vous l'avez dit, monsieur le ministre, la France ne peut pas être le terrain de jeu des trafiquants. De l'autre côté de l'Atlantique, la Guyane non plus ne peut pas être un territoire où tout est permis, où tous les moyens sont bons pour faire transiter de la drogue vers l'Europe.

détourner les contrôles renforcés que nous mettons en place. Nous avons bien évidemment sensibilisé la gendarmerie maritime pour prévenir de nouvelles tentatives de fraude de cette manière. Vous pouvez compter sur la détermination du Gouvernement pour lutter contre le trafic de stupéfiants en provenance de Guyane.

L'été est terminé et le bulletin de santé des services d'urgence est très inquiétant. Les faits sont là, abrupts. Dans nos départements, les plus ruraux en tête, ce sont des organes vitaux et structurants des territoires qui lâchent les uns après les autres. Dans les Alpes-de-Haute-Provence, mais la situation est similaire aux quatre coins de la France et des territoires d'outre-mer, l'organe vital des urgences de Sisteron est touché de plein fouet. Les urgences de nuit ont été suspendues cet été et n'ont pas rouvert depuis. Trois postes et demi manquent à l'appel. L'organe vital des urgences de Digne-les-Bains vient d'être touché à son tour. L'hôpital, qui assure 20 000 urgences par an, alors qu'un tel service est viable avec 12 000 patients, s'apprête à perdre quatre postes. Mêmes maux, mêmes constats pour l'organe des urgences de Manosque. Mes chers collègues, vous connaissez tous la chanson ! Or les médicaments et pratiques réanimatoires mobilisés ne produisent pas les effets escomptés. Je pense au recours massif aux sapeurs-pompiers et à la mutualisation des SAMU. Chacun sait, ici sur ces travées, que ce ne sont pas des solutions durables, humainement, écologiquement et financièrement. Alors oui, des recrutements sont prévus, mais les candidats ne se bousculent pas. Car comment les hôpitaux peuvent-ils rivaliser avec des structures privées qui s'arrêtent la nuit et sélectionnent les pathologies ? Comment rivaliser quand les services de biologie ou les plateaux techniques ne sont pas sur place ? Comment rivaliser avec des salaires faramineux en intérim de plus de 1 200 euros par jour qui flattent les comportements mercenaires ? Des mesures structurelles ont été prises. Mais, comme toute mesure structurelle, cela prendra du temps. Or du temps, nous n'en avons pas, parce qu'il s'agit de la vie et de la santé de nos administrés, mais aussi de la survie de nos territoires. Nous sommes tous des élus engagés au quotidien pour notre développement local, le numérique, les formations, le désenclavement, la lutte contre le réchauffement climatique. Comment pourrions-nous accepter que tout notre travail soit balayé d'un trait faute de médecins dans nos services d'urgence ? Madame la ministre, ma question est une proposition, car chaque territoire porte en lui ses solutions : quand organiserez-vous des Grenelles des urgences dans tous les départements ? Dans les Alpes-de-Haute-Provence, nous y sommes prêts maintenant

Nous pouvons et nous devons passer à l'action pour apporter aux Français une alternative concrète et attractive au « tout-urgences ». Nous devons créer, Mme la ministre l'a rappelé, le grand service d'accès aux soins qui manque à notre système de santé. Nous devons changer les modes de financement, aller plus loin et plus vite sur la reconnaissance et la valorisation

consigne au niveau national de fermeture des lits. Au contraire, nous devrons en ouvrir là où les besoins sont nécessaires et, surtout, en aval des urgences. La ministre a décidé de consacrer 750 millions d'euros au pacte de refondation des urgences,

pour trouver ensemble la réponse à ce problème de santé. Avec ces moyens, c'est tout le système Ma santé 2022 que nous complétons et que nous accélérons. La parole

vous avez annoncé renoncer à supprimer, dès l'an prochain, un avantage accordé jusqu'alors à toutes les personnes âgées de plus de 70 ans qui emploient une aide à domicile. Ce n'est pas de l'amateurisme de la part de votre gouvernement, mais le signe de votre déconnexion avec la réalité du quotidien de nos concitoyennes et concitoyens. Vous espériez ainsi piquer 300 millions d'euros dans les poches des retraités. Mais après la baisse de leur pouvoir d'achat à la suite de la hausse de la CSG et de la désindexation des pensions de retraite, leur colère vous a contraints à renoncer, et c'est tant mieux C'était le coup de trop à six mois des élections municipales pour votre majorité. Ma question est donc la suivante : maintenant que vous avez reculé sur les aides à domicile, quand allez-vous renoncer à votre réforme scélérate des retraites par points qui va en diminuer le montant ?

sous votre autorité, monsieur le président, ainsi que celle de nombreux sénateurs, je pense à Jean-Marie Vanlerenberghe, vous l'aviez déjà anticipé, notamment sur le système à points. Le regard que portent nos concitoyens sur le système actuel est sans ambiguïté. Ils le trouvent injuste, illisible, complexe, difficilement pilotable et surtout inadapté aux mobilités professionnelles nouvelles. La question de fond que nous nous sommes posée est la suivante : quel est le principe de base de la protection sociale du XXI siècle ? Comment garantir que l'avenir des retraites se fondera uniquement sur des solidarités professionnelles ? Nous offrons en réalité,

Vous refusez d'entendre la voix des milliers de personnes qui ont manifesté samedi dans de grandes manifestations. Vous refusez d'entendre la voix de ceux qui étaient dans la rue tout à l'heure. Nous étions, avec mes collègues du groupe CRCE, aux côtés de ces milliers de manifestants de manifestants que vous ne voulez pas entendre et qui remettent en cause le régime de retraite que vous leur présentez. Une société moderne doit accorder aux salariés le repos, et pour cela il faut qu'ils soient en bonne santé. Notre système de retraite universel par répartition garantit cela. Pour permettre à toutes et tous un départ à la retraite dès 60 ans, à 37,5 annuités, nous proposons de soumettre à contribution les 51 milliards d'euros de dividendes versés aux actionnaires au second semestre 2019 !

Que cherche-t-il en stigmatisant, il y a une semaine, de manière frontale, le droit d'asile dans notre pays ? Quel est ce préjugé qui voudrait que les classes populaires soient obligatoirement anti-migrants ? D'ailleurs, quelle est cette nouvelle division insidieuse que suggère le Président entre les catégories de Français, vision d'une nouvelle division, finalement, entre les Français ? Je vous interroge sur tout cela parce que nous ne comprenons pas où le Président veut nous emmener, si ce n'est vers des raccourcis contre lesquels il a été élu, dans un front républicain, en mai 2017. Nous ne comprenons pas non plus quel est le sens, en termes de santé publique, de la restriction voulue par l'exécutif sur l'aide médicale d'État, restriction d'accès qui cède à la plus grande démagogie, que j'ai malheureusement déjà entendue sur la droite de notre hémicycle. Enfin, et de manière plus circonstancielle, cette nouvelle offensive du Président sur les flux migratoires

Nous vous demandons des explications, monsieur le Premier ministre, car il est de plus en plus inquiétant que le Président tienne un double discours, qui dénonce les populismes et extrémismes au niveau international, tout en embrayant sur des idées différentes sur le plan national. Parler le langage de son adversaire, c'est un jour prendre le risque de le faire gagner. Alors oui, monsieur le Premier ministre, quel est ce jeu dans lequel vous voulez nous entraîner ? La parole est à M. le Premier ministre. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, monsieur le président Kanner, la semaine dernière, avec quelques membres du Gouvernement et les parlementaires de la majorité,

ce que l'on vous en a dit était incomplet. Il se trouve que j'étais présent, monsieur le président Kanner, et que j'ai entendu le discours du Président de la République : un discours d'une grande précision, d'une grande fermeté et d'une grande ouverture. Monsieur le président Kanner, j'ai indiqué, à l'occasion de ma déclaration de politique générale, que le Parlement, Assemblée nationale et Sénat, aurait l'occasion de discuter, discuter, fin septembre, début octobre, de la politique migratoire au sens le plus large pour notre pays, depuis les politiques d'aide publique au développement ou de coopération vers les pays d'origine jusqu'aux conditions d'intégrations des étrangers qui, venus en France, ont vocation à rester sur notre territoire, sans texte ni mesure. Très souvent, lorsque nous évoquons ce sujet, nous le faisons à partir d'un texte ou d'un ensemble de mesures, ce qui est parfaitement légitime, mais toujours un peu réducteur. L'objectif du Gouvernement, celui qui a été évoqué par le Président de la République, c'est que la représentation nationale puisse débattre, dans toutes ses dimensions, des questions que posent les migrations internationales, européennes, nationales, de l'amont à l'aval. premier point. Deuxième point : parler de l'immigration n'est pas un gros mot et n'est pas un petit sujet. Nos concitoyens en parlent, vivent cette question, ont des avis à formuler. Ils sont parfois divers, souvent contradictoires ; ils sont parfois empreints d'angoisse

méconnaître assez largement la réalité de l'opinion publique. Nous avons parfaitement le droit de ne pas être d'accord, vous et moi, mais j'ai le sentiment qu'évoquer de la façon la plus large possible ce sujet au sein de la représentation nationale n'est pas un contresens.

pour voir dans tous les domaines ce que nous pouvons faire, conformément aux principes qui nous guident, pour obtenir des résultats à la hauteur des enjeux. La parole Monsieur le Premier ministre, il n'y a pas d'angélisme de notre part, rassurez-vous, mais pas d'amalgame non plus. Nous serons toujours du côté de ceux qui pensent

et concerne le secteur de l'élevage, qui connaît de grandes difficultés, avec un prix de vente des bovins et ovins au niveau d'il y a vingt ans, non augmenté par la loi Égalim. Ma première question portera sur la sécheresse. L'agriculture devra, pour survivre, diversifier ses productions, avec la mise en place de retenues collinaires pour stocker l'eau de pluie afin de permettre l'abreuvage des animaux et l'irrigation des cultures. comment pourrait-on faciliter la procédure du stockage de l'eau, beaucoup trop longue, beaucoup trop complexe par rapport à d'autres États européens ? Enfin, quel bilan et quelles aides les pouvoirs publics peuvent-ils apporter cette année aux éleveurs victimes de sécheresse qui vont être obligés de vendre, de déstocker une partie de leurs animaux à un cours effondré ? Ma deuxième question concerne le CETA, signé le 30 octobre, partiellement appliqué avant la ratification des parlements. Celui-ci aura des effets bénéfiques pour certains secteurs, mais ce ne sera pas du tout le cas de l'élevage, notamment la viande bovine, puisque ce sont les règles de l'OMC qui s'appliquent et n'interdisent pas les farines animales pour l'élevage. Comment allez-vous appliquer l'article 44 de la loi Égalim, qui prévoit l'interdiction de proposer à la vente ou de distribuer à titre gratuit des produits importés pour lesquels il a été fait usage de produits vétérinaires ou d'aliments pour animaux interdits par la réglementation européenne ? Les éleveurs, inquiets, ont besoin de vous entendre de nouveau et d'être rassurés sur ce point.

Face à ce type de situation, l'objectif est de mobiliser le maximum d'herbe pour pouvoir la stocker, nourrir les animaux et éviter, comme vous l'avez dit, la décapitalisation. Le ministre de l'agriculture a ainsi immédiatement décidé d'activer les dérogations prévues pour les cas de force majeure. Cet été, soixante-neuf départements ont été concernés. Par ailleurs, pour redonner de la trésorerie aux éleveurs, le ministre a demandé à la Commission européenne une augmentation du taux d'avance des aides de la PAC. L'ensemble des mesures activables localement en cas de crise a été mobilisé pour redonner de la trésorerie aux agriculteurs exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, report ou allégement des cotisations versées à la Mutualité sociale agricole. Vous me permettrez en outre de saluer l'extraordinaire solidarité qui s'est exprimée une nouvelle

Il faut continuer à adapter nos pratiques pour réduire nos consommations et, surtout, rendre nos exploitations plus résilientes. Pour ce faire, les agriculteurs doivent avoir un accès sécurisé et facilité à l'eau. La France, reconnaissons-le, a accumulé un grand retard depuis des années sur ce sujet. Nous avons récemment débloqué la possibilité de construire des retenues collectives dans le cadre de projets de territoire. Les préfets ont pour mission désormais d'accompagner la réalisation des projets des agriculteurs, avec l'exigence de le faire dans des temps acceptables. concernant l'application de l'article 44 de la loi Égalim. Le CETA ne modifie aucunement les règles sanitaires applicables à l'entrée sur le marché européen. La réglementation européenne interdit l'importation de viande bovine issue d'animaux nourris avec des farines animales de ruminants et cette interdiction s'applique à tous les produits importés

Les agriculteurs sont les nouveaux boucs émissaires. Un suicide tous les deux jours, ce n'est plus tolérable ! La profession n'a pas attendu pour travailler à l'élaboration de chartes d'utilisation des produits phytosanitaires à proximité des habitations ou s'organiser ou s'organiser dans une démarche de responsabilité environnementale. Les agriculteurs connaissent les produits qu'ils utilisent ; ils ne vont pas traiter les jours où les enfants sont présents dans les écoles ou le dimanche à midi lorsque les familles déjeunent sur la terrasse. Ce sont des règles de bon sens. La mise en place de zones de non-traitement doit nous interpeller sur le principe même. Un produit dangereux à 3 mètres le sera tout autant à 10 ou à 150. Est-ce la distance ou la dangerosité du produit la source du problème ? La réduction de l'utilisation et la sortie des pesticides sont des enjeux environnementaux, économiques et sociaux importants pour l'avenir. Mais qui autorise la mise sur le marché ? Ce ne sont pas les agriculteurs Que l'on propose enfin des produits de substitution avec une innocuité avérée et une harmonisation européenne ! Les ZNT concernent à la fois l'agriculture conventionnelle et biologique. Je constate certaines incohérences. Comment atteindre les objectifs de surfaces agricoles en agriculture biologique si l'on supprime la possibilité d'utiliser les produits homologués bio tels que le cuivre, par exemple ? M. le ministre de l'agriculture l'a justement indiqué : des ZNT à plus de 100 mètres, c'est notre autonomie alimentaire qui serait mise à mal, avec plus de 20 % de surface agricole amputés et l'obligation de se fournir sur le marché mondial, avec des garanties sanitaires et environnementales moindres. Vous avez engagé une consultation. Gageons que le dialogue et la concertation dans nos territoires l'emporteront. Monsieur le Premier ministre, nous attendons votre réponse. La

sénateur Daniel Laurent, au nom de mon ministère, j'aimerais d'abord dire tout mon soutien aux agriculteurs qui vivent en ce moment des moments difficiles en matière d'agri-bashing. Vous avez rappelé les suicides des agriculteurs.

Ce travail, nous le menons avec les agriculteurs pour défendre toutes les agricultures en France : l'agriculture bio, l'agriculture de conservation des sols, les agricultures raisonnées et l'agriculture conventionnelle. La question des zones de non-traitement, les ZNT, est une question de protection des populations. La décision que nous avons prise avec le texte mis à la consultation est fondée sur l'avis de l'Anses, avis scientifique qui fixe entre 3 et 10 mètres les zones de non-traitement. Nous sommes bien loin des « coups de com » des maires prévoyant 150 mètres et qui voudraient rayer, du jour au lendemain, 20 % de la surface agricole utile. Néanmoins, nous avons besoin de ces zones de non-traitement pour prendre une mesure générale afin d'accompagner les dispositions figurant dans les autorisations de mise sur le marché, qui sont d'ailleurs parfois plus élevées en fonction de la nature du produit La consultation nous permettra d'avancer sur ce sujet.

portant création de la métropole Aix-Marseille-Provence, ou AMP, a prévu de doter ce nouvel établissement public de coopération intercommunale de plusieurs compétences dites « de proximité Le transfert de la compétence « voirie communale » devait initialement être mis en oeuvre avant le 1 janvier 2018. La loi relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain du 28 février 2017 a finalement repoussé cette échéance au 1 janvier prochain. Depuis ce report, le débat sur l'avenir de la métropole AMP s'est poursuivi. M. le Premier ministre a demandé l'an passé au préfet de région de conduire une mission de concertation sur les mutations possibles de l'actuel EPCI. Dans cette perspective, un dialogue a été établi établi avec les élus locaux et un rapport a été remis au Gouvernement. Ces échanges et les travaux conduits par M. le préfet font apparaître une préoccupation commune de voir la métropole se concentrer sur les projets les plus structurants de son territoire tout en renvoyant l'exercice de certaines compétences de proximité, notamment la voirie, vers les communes, au plus près du terrain. Un transfert au 1 janvier 2020 des compétences « création, aménagement et entretien de voirie » et « création, aménagement et entretien des espaces publics dédiés à tout mode de déplacement urbain ainsi qu'à leurs ouvrages accessoires » n'apparaît plus opportun au moment où une réflexion nouvelle est engagée sur la répartition des rôles entre communes et métropole dans les Bouches-du-Rhône. Aussi, monsieur le ministre, dans l'attente des propositions de l'exécutif sur le devenir de la métropole AMP, le Gouvernement serait-il favorable à une annulation ou à un nouveau report du transfert de ces compétences

de la loi Maptam et le calendrier tel que le législateur l'avait imaginé. Soyons pragmatiques : le transfert de la compétence « voirie » peut-il se faire dans de bonnes conditions au 1 janvier 2020 ? Si l'on écoute l'ensemble des acteurs du territoire, la réponse est non.

Ma question s'adresse à M. le ministre de l'économie et des finances. Monsieur le ministre, Thomas Cook, le plus vieux voyagiste au monde, vient de déposer le bilan, laissant 600 000 voyageurs en attente de rapatriement, dont 10 000 Français. Mais c'est aussi et surtout tout un ensemble de prestataires qui se trouve aujourd'hui dans une situation périlleuse : hôteliers, restaurateurs, autocaristes, organisateurs de spectacles, de croisières. En métropole, aux Antilles, en Corse, pas moins de 2 000 locations touristiques, plusieurs centaines d'hôtels, près de 200 croisières, 500 clubs de vacances et campings Monsieur le ministre, à court terme, la promesse de Thomas Cook est d'indemniser l'ensemble de ses clients, mais qu'en est-il de ses prestataires, auxquels Thomas Cook n'aura rien versé et qui sont dans l'incapacité de revendre leurs prestations dans un délai très court ? Je vous rappelle que les PME du secteur du tourisme sont déjà dans une situation économique tendue après les mois de violences en marge des manifestations des « gilets jaunes », lesquelles ont provoqué des pertes de chiffre d'affaires importantes et non indemnisables. À moyen terme, quel va être l'avenir des quelque 400 agences Thomas Cook en France, filiales en propre ou franchisées ? Enfin, à long terme, monsieur le ministre, n'assistons-nous pas, par la faillite de Thomas Cook, à un phénomène beaucoup plus large d'effondrement du modèle économique des agences de voyages physiques au profit d'un modèle dématérialisé, où seuls les géants comme Expedia, Booking ou Google pourront subsister ? La parole est

votre question porte sur la situation de Thomas Cook, placé hier en situation de liquidation judiciaire. Comme vous l'avez dit, cette affaire pose le problème de la fragilité de certains opérateurs du secteur touristique face à une concurrence intense et à la montée des plateformes numériques. S'agissant précisément de la situation des 10 000 Français

Je veux donc vous rassurer sur la situation de nos compatriotes et vous dire aussi que les Français sont bien protégés dans le secteur du tourisme, non seulement par le mécanisme français dit « APST », mais aussi par le système de garantie européen.

les 780 emplois français touchés par cette mesure, le Gouvernement est en liaison avec la direction de Thomas Cook France et prendra les mesures de soutien adaptées. Là aussi, vous pouvez compter sur notre vigilance et notre action. La parole

Madame la ministre, après la hausse de la CSG, après la décision de ne plus indexer les retraites sur le coût de la vie, avant une réforme des retraites qui réduira inévitablement le niveau des pensions et creusera les inégalités, le Gouvernement comptait s'attaquer de nouveau aux personnes âgées en ciblant, cette fois, l'exonération de charges sociales dont bénéficient les plus de 70 ans employant une aide à domicile. Encore un mauvais coup porté à leur pouvoir d'achat Or nous venons d'apprendre que le Gouvernement renonçait à cette mesure, qui devait pénaliser près de 800 000 bénéficiaires. Face à l'émoi suscité par une décision injuste prise sans concertation, constatant une fois de plus que la méthode n'est pas la bonne- bonne- le Premier ministre l'a reconnu lui-même à l'Assemblée nationale cet après-midi -, l'exécutif a été contraint de reculer. À deux jours de la présentation du budget, veille du conseil des ministres, vous êtes dans l'improvisation la plus totale ! Pour autant, d'autres mesures d'économies annoncées dans le prochain budget 2020 sont particulièrement inquiétantes.

un chômeur sur deux verra son allocation baisser ! Aussi, madame la ministre, ma question est simple : pouvez-vous vous engager, sur ces mesures profondément injustes, à revoir votre copie, en privilégiant cette fois la concertation et le dialogue social ?

pour l'assurance chômage : aucun demandeur d'emploi ne verra son capital de droits diminuer. Simplement, ceux qui gagnaient provisoirement plus au chômage qu'en travaillant

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, ma question porte sur la circulaire dite « zéro artificialisation nette », parue dans l'été, invitant les préfets à la fermeté à l'égard des documents d'urbanisme. Tant sur le fond que sur la forme, il ne souffle pas vraiment un esprit de décentralisation dans ce texte. Alors que le dialogue entre les élus des territoires et le Gouvernement s'était réchauffé, cette circulaire signée par quatre ministres le refroidit sérieusement. Si la sobriété de la consommation foncière, dont la lutte contre l'artificialisation, est un objectif réel et louable et, j'ose le dire, partagé, en revanche, la méthode proposée jette l'opprobre sur les élus locaux, les rendant suspects d'une inconscience coupable. Que les préfets et l'État accompagnent la rédaction des documents d'urbanisme, c'est légitime, et même souhaitable. Ces échanges dans le respect sont indispensables. Mais, en l'occurrence, si le document approuvé va à l'encontre « de l'objectif affiché il est demandé aux préfets de « mobiliser tout l'éventail de leviers réglementaires », qui va de l'avis défavorable jusqu'à la suspension du caractère exécutoire du document. Les élus concertent et dialoguent avec l'État, décident ensemble, en conscience, d'un document d'urbanisme qu'ils votent, mais l'État peut tout bloquer. Sur quels critères Que pèse donc le vote par des élus d'un SCOT aux yeux de l'État ? Où est l'autonomie des collectivités ? Vous le savez, les territoires qui vont en pâtir sont ceux-là mêmes qui voient les services partir, la poste, les écoles fermer, leur population vieillir Pour quelques territoires jugés déraisonnables, on décide de léser tous les autres. Monsieur le ministre, les mots ont un sens en ces temps de dialogue affiché. Attendre des préfets qu'ils provoquent « une prise de conscience et une modification des comportements », c'est leur prêter bien plus qu'un rôle réglementaire, vous en conviendrez, et c'est vexatoire. Les territoires sont inquiets ! Comment comptez-vous les rassurer et garantir à une petite commune rurale qu'elle a un avenir dans la République ?

Dans la suite de la discussion générale, la parole est à M. Frédéric Marchand. Monsieur Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, l'examen du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire intervient dans un contexte d'urgence qui nous impose, collectivement, d'être à la hauteur des enjeux. Nous démarrons ainsi cet examen quatre ans après que 193 pays ont décidé, le 25 septembre 2014 à l'ONU, d'embarquer ensemble sur la voie du développement durable, pour « se se consacrer collectivement à la poursuite du développement mondial et d'une coopération mutuellement bénéfique, susceptibles d'apporter d'énormes gains à tous les pays et toutes les régions du monde Parmi les points figurant à cet agenda 2030, l'objectif 12 est celui qui retient toute notre attention, avec une volonté affichée d'aller vers une consommation et une production responsables. Aujourd'hui, nos concitoyens nous disent qu'il y a urgence à réfléchir et agir pour les producteurs, les consommateurs et les autorités publiques sur nos habitudes, nos usages en termes de consommation, de production de déchets l'impact environnemental et social de l'ensemble de la chaîne de valeur de nos produits. Oui, madame la secrétaire d'État, sur un sujet essentiel pour notre avenir collectif, vous avez fait le choix de la concertation la plus large qui soit, associant entreprises, associations, collectivités et experts, sans oublier plus de 5 000 contributions publiques. C'est un véritable projet de société conçu dans cette feuille de route qui enclenche la transition d'une économie linéaire, basée sur le modèle « fabriquer, consommer, jeter », vers une économie circulaire, une économie différente où nous consommons de manière sobre, où les produits ont une durée de vie plus longue, où nous limitons les gaspillages et où nous arrivons à faire de nos déchets de nouvelles ressources. Notre commission s'est pleinement saisie du sujet, dans un calendrier certes contraint, mais avec une forte appétence et un souci partagé : donner à ce texte tous les moyens de ses ambitions pour en faire un texte de référence. Notre rapporteure, Marta de Cidrac, a multiplié les auditions pour nous permettre de mieux appréhender les problématiques et de sortir d'une vision parfois trop « techniciste » sur certains sujets, comme celui des déchets, pour basculer vers une dimension politique et sociétale. Les sujets de convergence entre nous sont nombreux, notamment s'agissant de l'information qui doit être donnée au consommateur pour qu'il devienne véritablement éco-responsable. Nous pouvons sans doute aller plus loin en matière de lutte contre le gaspillage, de durabilité et de réparabilité. Notre groupe fera des propositions en ce sens.

La question de la responsabilité élargie du producteur, ou REP, est aussi au coeur de ce projet de loi. Déployée depuis vingt-cinq ans, elle a considérablement contribué au développement du recyclage dans notre pays, mais il lui faut désormais aller plus loin, au travers de la création de nouvelles filières, mais aussi, et surtout, en arrêtant le principe d'une responsabilité universelle du producteur l'amenant à s'interroger le plus en amont possible sur la gestion de ses produits en fin de vie. J'aimerais aussi évoquer avec vous la situation de nos territoires ultramarins. Ces derniers font face à un retard important en matière de traitement des déchets. Les raisons sont multiples, mais tiennent principalement à un manque d'infrastructures notoire et à un désintérêt évident des éco-organismes. Nous devons agir au plus vite afin de mieux organiser le déploiement effectif des REP sur ces territoires et d'encourager le développement d'une coopération par bassin qui permette d'atteindre la masse de déchets suffisante pour créer des filières efficaces et rentables. Par ailleurs, nous ne pouvons pas nous contenter du statu quo. La création d'une instance de suivi et d'observation des filières REP, en liaison avec l'Ademe, avec des moyens dédiés, est sans doute une priorité sur laquelle nous devrons de nouveau travailler. Évoquer les nouvelles filières, c'est aussi s'arrêter quelques instants sur l'épineuse question des déchets du bâtiment. L'amélioration de la gestion de ces derniers et la lutte contre les dépôts sauvages sont au coeur de nos débats. Nous pouvons certainement pousser plus loin les curseurs en liaison avec les acteurs de la profession. Démontabilité, réemployabilité, séparabilité, recyclabilité sont des paramètres sur lesquels il convient d'avancer à marche forcée, tout comme sur certains secteurs comme le verre, le plâtre, les sols souples et les parquets. Nous devons nous interroger sur la question de la transformation sur site des déchets ou bien encore sur le lancement d'un grand plan de recherche et développement pour l'économie circulaire dans le BTP. Je n'oublie pas non plus le rôle des éco-organismes, au coeur de nos préoccupations, et nous nous rejoignons quand nous disons qu'il faut à la fois repenser leurs missions et leur gouvernance. Il semble essentiel par exemple que l'éco-conception, l'intégration des matières recyclées entrent dans leur champ. Nous le voyons bien, ce texte, n'en déplaise à ses contempteurs, s'inscrit dans la dynamique de transition écologique à laquelle s'est attelé le Gouvernement. Il pose les bases d'un nouveau modèle de société en inscrivant notre pays dans une vision collective européenne. Comme me le faisaient remarquer les élus du Syndicat mixte intercommunal de collecte et de valorisation du Libournais Haute-Gironde, avec qui ma collègue Françoise Cartron et moi-même avons eu l'occasion d'échanger, ce projet de loi décline un « nouveau cadre législatif ambitieux et offensif ». Alors oui, l'ambition et l'offensive de ce texte ne se résument pas à la seule question de la consigne pour recyclage des bouteilles en plastique. Notre commission a revu le texte en se consacrant sur la consigne pour réemploi et réutilisation, sujets aujourd'hui prioritaires. Pour autant, il serait irresponsable d'écarter d'un revers de main la question du recyclage du PET. Le sujet mérite qu'on s'y arrête de manière sereine, en intégrant tous les paramètres d'un système à la française unique en son genre, notamment en raison de la place des collectivités dans le dispositif. Au-delà, c'est toute la question de la place du plastique dans notre vie quotidienne qui est posée et il me paraît donc, à ce stade de nos discussions, que nous ne devons pas confondre vitesse et précipitation. Mais nous aurons sans doute l'occasion, les uns et les autres, de nous exprimer dans le cadre de l'article 8. Madame la secrétaire d'État, nous partageons toutes et tous avec vous l'ambition de changer de paradigme. Vous pouvez compter sur le groupe La République En Marche pour contribuer activement à la mise en oeuvre de ce nouveau modèle que nous appelons tous de nos voeux. La parole

En effet, il est plus que temps, pour reprendre vos mots, madame la secrétaire d'État, de changer de paradigme. Recycler est un point de départ indispensable, mais pas une fin en soi. Le défi de notre économie est de réduire drastiquement sa production de déchets. Dès la conception du produit, il faut penser à la fin de sa première vie. Dès le choix des matériaux et de leur assemblage, tout doit être pensé réparable, réutilisable, réellement biodégradable ou, au pire, recyclable. Il faut passer de l'ère du jetable à l'ère du durable. Cela implique de sortir du productivisme et du culte de la croissance coûte que coûte, incompatible avec ce concept. Cela implique une révolution de notre modèle économique que ce projet de loi n'effleure qu'à peine. Notons néanmoins que ce texte comporte des avancées intéressantes. L'information simplifiée des consommateurs est bienvenue. La création de nouvelles filières REP pour améliorer la collecte de nombreux déchets problématiques comme les piles, les mégots

Tout cela va dans le bon sens, mais reste largement insuffisant. Comme pour la loi d'orientation des mobilités, nous sommes face à un texte sympathique, nourri de bonnes intentions, mais qui ne répond concrètement que très partiellement à l'urgence écologique. Alors, madame la secrétaire d'État, vous communiquez intelligemment sur le retour de la consigne, que tout le monde souhaite.

en cherchant à lui donner une image plus vertueuse, un système économique que nous devons faire disparaître ! Ce faisant, selon une vilaine habitude bien connue- la privatisation des profits et la socialisation des pertes -, le secteur privé cherche à mettre la main sur la partie la plus rentable de la gestion des déchets- le recyclage des bouteilles en PET laissant à la charge des collectivités et des contribuables tout ce qui ne rapporte pas d'argent. Avouez que la ficelle est un peu grosse ! Je ne m'étends pas plus sur ce sujet, qui occupera nombre d'heures durant nos débats, mais j'en profite pour saluer les modifications introduites en commission sur l'initiative de plusieurs groupes, notamment

l'avons fait pour vous ... -, cela ne réglerait en fait pas grand-chose ! Fabriquer une bouteille plastique nécessitera toujours 70 % de résine neuve. L'économie du plastique n'est pas circulaire, et on ne voit vraiment pas comment elle pourrait le devenir. On parle ici, rappelons-le, d'un produit pétrolier, donc d'une ressource non renouvelable, qui se dégrade très lentement et pollue chaque recoin de la planète, même le coeur du Pacifique. On parle d'objets, le plus souvent à usage unique, qui sont brûlés, ce qui rejette près d'un milliard de tonnes de CO2 chaque année. On parle d'un produit que nous n'arrivons même pas à recycler chez nous, tant nous produisons de déchets, et que nous envoyons au fin fond de l'Asie, où il n'est que partiellement recyclé et s'accumule dans les décharges chinoises ou malaisiennes, pays qui ferment un à un leurs portes à nos cargos, car ils en ont assez- c'est légitime -de nous servir de poubelles. Madame la secrétaire d'État, il faut arrêter les frais tout de suite ou l'humanité finira ensevelie sous ses déchets plastiques. Or votre projet de loi ne propose pas de scénario de sortie du plastique ni de mesures pour réduire à la source son usage. Rien sur la vente en vrac, pas grand-chose sur le suremballage, ce texte manque cruellement de signaux forts Ce matin, vous invitiez Greta Thunberg « à sortir de l'incantation » et à proposer des solutions. Nous ne résistons pas à l'envie de vous retourner le compliment. Vos solutions demeurent très éloignées de l'ambition affichée du projet de loi, qui, du coup, semble quelque peu incantatoire. Comme toujours, l'ambition écologique du gouvernement auquel vous appartenez s'arrête quand elle rencontre les intérêts des industriels. Avec ce boulet au pied, vous ne pouvez pas avancer : les intérêts de Coca-Cola et ceux des tortues ou des goélands ne sont pas compatibles ; les intérêts de Pepsi et ceux de la civilisation humaine non plus ! Nous savons que vous faites des efforts pour convaincre un Premier ministre rétif. Nous savons que vous êtes contrainte par les équilibres gouvernementaux, qui vous brident. Aussi, nous vous proposons notre aide. Nous vous proposons de donner un cadre légal à la vente sans emballage ni gâchis pour amplifier l'effort citoyen qui Nous vous proposons une trajectoire de sortie du plastique jetable d'ici à 2040. Nous vous proposons de standardiser les contenants en verre pour créer une vraie consigne digne de ce nom. Nous vous proposons d'apprendre aux enfants à réparer plutôt que de devoir jeter. Nous vous proposons d'étendre les délais de garantie des objets. Nous vous proposons d'enrichir la formation des architectes pour réduire à la source le gisement colossal des déchets du secteur de la construction. Nous vous proposons des objectifs, notamment en termes de commande publique, et des moyens pour dynamiser le secteur du réemploi solidaire, qui redonne vie à nos objets. Nous vous proposons un arsenal pour lutter contre l'obsolescence logicielle sournoise, fléau du secteur électronique. Nous mettons sur la table, sous vos yeux, une myriade de solutions imaginées par les actrices et les acteurs de l'économie circulaire, qui n'ont pas attendu ce projet de loi pour passer de la culture du jetable à celle du durable ; une myriade de solutions pour faire de votre texte la grande loi du XXI siècle qu'il mérite d'être.

nous avons pu faire adopter notre amendement de manière quasi unanime et ne pas acter une consigne sur les bouteilles plastiques écrite par et pour les industriels de la boisson. Espérons que cette consigne, qui n'a rien à voir avec le souvenir de la consigne du verre que nos anciens ont connue, ne revienne pas par la fenêtre ! Malgré le bel emballement et, si j'ose dire, l'emballage médiatique de la consigne que le Gouvernement tend à vendre aux Français, le Sénat s'est courageusement élevé contre cette mesure inique qui consiste à privatiser une nouvelle fois une part du service public assuré par les collectivités locales. s'agissait bien de cela ! L'objectif avoué du Gouvernement est bien, sous couvert d'atteindre un taux de recyclage de 90 % des seules bouteilles plastiques en PET clair, d'instaurer une consigne qui obligerait les citoyens à ne plus utiliser leur bac jaune, mais à remettre ces bouteilles contre rémunération dans des automates gérés par le secteur privé.

est un indice de la proximité qui existe entre vos services et le collectif Boissons- la presse spécialisée s'en est fait l'écho. Cette proximité avec les lobbies a déjà fait fuir un certain Nicolas Hulot Il faut que les Français comprennent les raisons profondes qui nous animent, car nous partageons les objectifs de réduction du plastique. Le sujet est plus complexe qu'il n'y paraît. Ce projet de consigne a tout de la fausse bonne idée. Premièrement, notre système de gestion et de traitement des déchets est actuellement en pleine refonte en raison de la généralisation des consignes de tri. Cette grande transformation, qui engage plusieurs milliards d'euros d'investissements de la part des collectivités, va permettre à la France de se doter d'un outil public extrêmement performant

C'est une révolution silencieuse qui est déjà bien enclenchée. Les exemples de la Belgique ou de la Suisse sont là pour nous confirmer que ce système de gestion publique des déchets peut tout à fait fonctionner sans consigne pour recyclage. l'objectif de 90 % est à portée de main pour les collectivités, et c'est de la chambre des territoires que nous vous adressons ce message ! De plus, avec ce système, ce n'est pas 90 % que les collectivités vous proposent d'atteindre, mais 100 % des emballages plastiques recyclés d'ici à trois ans, ce qui correspond d'ailleurs à l'un des engagements du Deuxièmement, le modèle français de gestion des déchets tire sa force de la simplicité du geste de tri et de la collecte en porte-à-porte. Demander aujourd'hui aux Français de changer leurs habitudes de tri, et uniquement pour certains emballages comme les bouteilles plastiques, est un non-sens et risque, ce qui est confirmé par une étude de l'Ademe sur le sujet, de perturber les efforts réalisés sur d'autres catégories de déchets. Si la consigne était un système miracle, cela se saurait ! De nombreuses études illustrent le fait que sa mise en place n'a aucun impact sur la réduction des déchets sauvages ou sur la consommation de plastique à usage unique. Ainsi, en Allemagne, la consigne a provoqué une explosion de la consommation des bouteilles en plastique. Le système de consigne pour recyclage valide en réalité la consommation de plastique, en déculpabilisant l'acte d'achat. Le consommateur-citoyen se voit rassuré et encouragé à acheter des bouteilles en plastique plutôt que de s'interroger sur leur prolifération. Vous le savez, cette consigne est conçue par et pour les vendeurs de boissons. Et voilà qu'hier vous déposez en catastrophe un amendement pour sauver ce dispositif promis à un avenir incertain dans cet hémicycle Nous y reviendrons dans le débat, mais j'attends toujours la réponse à ma question : quelle est la plus-value pour le citoyen qui d'ores et déjà mettait sa bouteille plastique dans le bac jaune ? Et je ne parle même pas des collectivités, qui vont devoir faire le tri entre les bouteilles consignées et celles qui ne Quelle usine à gaz ! Quelle impréparation ! Est-ce comme cela que vous envisagez la concertation avec les collectivités territoriales ? Permettez-moi de dire qu'on tourne en rond ! En dernier lieu, j'aimerais insister sur un point qui nous est cher le sujet de ce projet de loi est-il de savoir si l'on est pour ou contre la consigne ou bien est-ce de trouver les moyens de sortir de cette civilisation du plastique Vous le savez, le plastique est aujourd'hui le premier débouché de l'industrie pétrochimique. Ce n'est pas simplement aux citoyens de changer leurs comportements, mais bien aux metteurs en marché de repenser leur surutilisation. Le plastique se retrouve partout et représente une pollution massive qui s'introduit dans l'air, dans l'eau- jusqu'au fond des océans -et dans les sols. Toutes les études scientifiques démontrent que l'anthropocène a pour autre nom « plasticocène », l'ère du plastique. Devant ce fléau massif qui s'observe aussi bien à l'oeil nu qu'au microscope, nous proposons de nombreuses mesures de lutte contre cette pollution. Nous pensons que là est le vrai débat de ce texte, et vos discours, madame la secrétaire d'État, tendent à nous convaincre que vous n'êtes pas loin de partager ce point de vue. Ne prenons pas ce sujet par le petit bout de la lorgnette- la consigne sur les bouteilles plastiques mais élargissons ce combat à l'ensemble des emballages et des plastiques à usage unique ! Parlons des microfibres synthétiques qui se retrouvent dans nos rivières et que les stations d'épuration sont dans l'impossibilité de filtrer. Parlons du suremballage des aliments et des produits. Parlons de la hiérarchie des modes de traitement du déchet. Parlons du recyclage des plastiques consommés hors foyer. Donnons ensemble des objectifs clairs et chiffrés à nos entreprises pour qu'elles s'engagent dans une transition circulaire. Parlons de l'obsolescence programmée de nos biens dits durables. Parlons réemploi et export de nos déchets. Voilà la forêt de plastique cachée par la consigne sur les bouteilles ! Les Français nous attendent sur tous ces sujets pour dessiner l'écologie, non pas de demain, mais d'aujourd'hui.

À ce titre, l'un de nos premiers amendements vise à prévoir un grand plan national de lutte contre la pollution plastique à partir de 2020. La France, en tant que premier producteur européen de déchets plastiques, a une responsabilité importante. Au regard Au regard de la pénétration profonde de cette matière dans la totalité de nos écosystèmes, il est urgent de se doter d'un cadre juridique pour réduire efficacement la production et la consommation de plastique, en se donnant des objectifs contraignants. Par ailleurs, si vous ne vous étiez pas braquée sur cette consigne, nous aurions pu, sincèrement, accueillir votre projet de loi avec bienveillance, car de nombreuses dispositions nous semblent intéressantes, tout en méritant C'est le cas du renforcement de l'information aux consommateurs, qui est prévu au titre I et qui nous semble crucial pour développer l'économie de la réparation et du réemploi, économie très présente sur nos territoires. À titre d'exemple, les ressourceries affichent chaque année des records de fréquentation et ont impulsé une économie du réemploi, du don et de la réparation. Je pense aussi à la réussite des territoires « zéro chômeur de longue durée », lancés sous la précédente législature et qui, grâce au soutien de l'économie sociale et solidaire, permettent de ranimer des territoires ruraux et de redonner de l'espoir aux citoyens privés d'emploi. En ce sens, il est très important de créer le fonds de réemploi solidaire pour booster ce secteur économique. Le succès remporté par les applications d'aide à l'achat responsable démontre aussi, à bien des égards, l'intérêt des Français pour connaître la qualité des produits, leur traçabilité ou encore leur impact écologique. Il apparaît essentiel de rendre aux consommateurs-citoyens l'information qui leur est due. Si nous voulons véritablement changer nos modes de consommation en sorte que le marché se plie à l'impératif environnemental, l'information est un levier redoutable et très efficace. En outre, la lutte contre les invendus non alimentaires prévue à l'article 5 emporte également notre adhésion. très impliquée, madame la secrétaire d'État, sur ce thème depuis la destruction d'invendus par Amazon et encore récemment par Go Sport, mais pour qu'un souhait se réalise, il faut assortir cette velléité de sanctions efficaces, ce que nous proposerons. Il faut également faciliter le don, en rectifiant des aberrations fiscales qui encouragent les entreprises à détruire leurs invendus plutôt qu'à les donner à des associations. Autre point largement positif : la création de nouvelles filières de responsabilité élargie des producteurs, les REP, prenant en charge des déchets jusqu'ici destinés à l'incinération ou à l'enfouissement faute de possibilité de recyclage. La refonte du fonctionnement des éco-organismes est également fondamentale. Enfin, nous vous soutenons dans la mise en place d'une REP dans le secteur du bâtiment, qui pourrait être une solution pour mettre fin au scandale des déchets sauvages vécu par d'innombrables citoyens et élus locaux qui luttent parfois au péril de leur vie contre ce désastre écologique. Se pencher sur l'économie circulaire, c'est donc s'interroger profondément sur le système de production. C'est prendre en compte la totalité du cycle de vie d'un produit créé. C'est, en un mot, devenir responsable. C'est l'introduction de la rationalité écologique dans la rationalité économique. Moins de ressources, mais une meilleure conception pour favoriser une économie de la fonctionnalité. C'est tout le sens de l'éco-conception à la base des produits qui sont mis sur le marché, à laquelle nous sommes très attachés. Vous l'aurez compris, madame la secrétaire d'État, nous sommes loin de nous opposer de manière dogmatique à ce projet de loi- bien au contraire Toutefois, il faut arrêter de vouloir cornériser les parlementaires, en l'occurrence les sénateurs, qui sont à l'écoute des territoires et connaissent bien la question de la gestion et du traitement des déchets. Il aurait été judicieux de lancer une véritable concertation avec ceux qui détiennent l'expertise plutôt qu'avec des industriels attirés par le gain. Malgré votre campagne de communication agressive à l'égard d'un Sénat qui serait rétrograde en matière environnementale, nous vous tendons la main et vous demandons de bien vouloir entendre les représentants des territoires. La parole

En effet, le gaspillage est intolérable, tout le monde en conviendra. Quant au passage d'une économie linéaire à une économie circulaire, elle est la condition pour que notre civilisation perdure. Mais passé l'intitulé du texte, les choses se corsent ... Notre commission de l'aménagement du territoire et du développement durable a émis un avis très sévère sur le projet de loi. Je dois dire, madame la secrétaire d'État, que nous le partageons : sorti de la transposition des directives, de l'élévation au rang législatif de mesures réglementaires qui figuraient déjà dans la feuille de route pour l'économie circulaire et des fameuses habilitations à légiférer par ordonnance, le texte nous paraissait très en retrait par rapport à ce que nous pouvions en attendre. Pis, la fameuse consigne sur les bouteilles en plastique, pourtant présentée comme la mesure phare du projet ... Je ne l'ai jamais présentée ainsi ! ... est un non-sens écologique. Alors, parlons de cette consigne pour purger la question. Je commencerai par une petite mise en perspective : il est amusant de constater que cette mesure a polarisé les esprits et risque d'occuper une bonne partie de la discussion parlementaire, alors même que les bouteilles en plastique ne représentent que 0,2 % de l'ensemble des déchets générés en France chaque année. Il est vrai que la pollution du plastique, à laquelle les bouteilles participent largement, est l'une des plus graves qui soit. Toutefois, il faut admettre que le sujet de l'économie circulaire est autrement plus vaste. On ne compte plus les arguments contre l'instauration de cette consigne. Premièrement, elle est décidée par le Gouvernement sans véritable concertation. En audition, les responsables de l'Ademe, organisme auquel incombe institutionnellement l'évaluation de tels dispositifs, se sont dits incapables de se prononcer aujourd'hui sur ce sujet ; il leur faut plus de temps. Deuxièmement, nous avons de bonnes raisons de penser que l'instauration d'une consigne sur les bouteilles en plastique n'est pas indispensable pour atteindre l'objectif européen de 90 % de bouteilles de bouteilles recyclées en 2025. C'est ce que révèle le rapport Stefanini commandé cet été par la commission du développement durable. Quand on ne prend en compte que ce qui est collecté auprès des ménages, les taux actuels de recyclage sont bons et progressent De plus, la marge d'amélioration sur la collecte hors foyer est importante. À ce niveau, je voudrais également évoquer une disposition du Grenelle qui, une fois mise en oeuvre, donne d'excellents résultats au niveau de la collecte de la tarification incitative, plus particulièrement de la redevance incitative. Troisièmement, la consigne est une mauvaise nouvelle pour le consommateur. Aujourd'hui, il paye sa bouteille à un prix donné et, quand elle est vide, il la jette en bas de chez lui dans le bac approprié. Simple, basique ! Demain, avec la consigne, il devra la payer plus cher et la rapporter au magasin. Madame la secrétaire d'État, vous vous prévalez du soutien de l'opinion publique pour défendre la consigne ; il suffit pourtant d'expliquer cela aux gens pour qu'ils changent d'avis.

et un cadeau direct, si la consigne ne fonctionne pas autant qu'espéré, car toute bouteille qui ne sera pas rapportée fera gagner au metteur en marché le montant de la consigne correspondante. Pendant ce temps-là, les collectivités auront investi à perte. C'est le cinquième argument. Alors que les collectivités sont incitées à moderniser le tri depuis des décennies et qu'elles ont déjà réalisé la moitié des investissements nécessaires, on leur impose, du jour au lendemain, un virage à 180 degrés. En termes de sécurité juridique et de confiance légitime, c'est un cas d'école ! Le résultat, c'est que les collectivités ont gelé tout nouvel investissement depuis l'annonce de la mise en place de la consigne. Elles ont raison, puisque, si la consigne est créée, les investissements déjà réalisés l'auront été à perte. La matière qui a de la valeur va se retrouver aux mains des industriels, tandis que ne restera plus au service public des déchets La perte non compensée pour les collectivités serait de 240 millions d'euros par an en 2022, alors même qu'il leur faudra mettre en place l'extension de la consigne de tri à tout emballage et, en 2025, la gestion des biodéchets. Le dernier argument, le sixième, est le plus important. S'il ne fallait en retenir qu'un, ce serait celui-là : la consigne est un non-sens écologique ! Dans sa version initiale, il s'agissait d'une consigne pour recyclage. Or, on le sait, dans la hiérarchie des modes de traitement des déchets, le recyclage n'arrive qu'en cinquième place. Avant d'envisager le recyclage, il faut tâcher de diminuer le volume des déchets et penser à la réparation, à la réutilisation et au réemploi. Si rien de tout cela n'est possible, alors oui, le recyclage devient un mode de traitement. En l'occurrence, recycler le plastique signifie produire toujours plus de plastique. Car, quand une bouteille est faite avec 30 % de plastique recyclé, cela signifie qu'il a fallu fabriquer 70 % de plastique nouveau C'est un cercle vicieux. Tous les pays qui ont adopté un tel système, à commencer par l'Allemagne, pays que je connais bien, ont vu la part du plastique monter en flèche sur leur marché. C'est bien pourquoi, comme notre rapporteure, nous avons déposé en commission un amendement visant à limiter le principe de la consigne à la réutilisation et au réemploi, ce qui, pour le coup, est vraiment écolo ! Nous ne pouvons que nous en féliciter. De même, nous approuvons les autres améliorations apportées au reste du texte par nos rapporteures : Marta de Cidrac, saisie au fond, et ma collègue du groupe UC Anne-Catherine Loisier, saisie pour avis. Je les félicite pour l'excellence de leur travail. Nous saluons les efforts de simplification faits dans le cadre de l'information du consommateur, mais l'apport le plus considérable du Sénat est la valorisation, dans tous les aspects du texte, des modes prioritaires de traitement des déchets valorisation de la réduction du volume de déchets par la fixation d'objectifs de lutte contre le suremballage ; valorisation de la réparation par la création d'un fonds dédié à ce mode de traitement au sein des éco-organismes ; valorisation du réusage et du réemploi dans tous les achats publics ou par le recentrage de la fameuse consigne. La commission a aussi effectué un gros travail de refonte du cadre applicable aux éco-organismes, en réformant leur régime de sanction et en leur fixant des objectifs distincts de réduction des déchets, de réemploi et de recyclage. Le groupe UC a pris sa part à cette refonte, en faisant adopter un amendement qui élargit la gouvernance des éco-organismes à toutes les parties prenantes. Chacun le sait, les éco-organismes sont insuffisamment contrôlés. Le nouveau texte devrait remédier De même, nous nous félicitons de l'adoption de notre amendement qui généralise le recours à l'éco-modulation afin de faciliter l'atteinte des objectifs fixés aux éco-organismes. des modes de traitement des déchets, la commission et le groupe UC ont aussi oeuvré à privilégier la valorisation énergétique pour réduire au maximum le recours au stockage. C'est toute la problématique du développement des combustibles solides de récupération. Je salue enfin l'effort fourni pour lutter contre les dépôts sauvages. Le Sénat a joué son rôle, en lui consacrant un titre nouveau dans le texte. Le groupe UC pense qu'il faut aller encore plus loin, en renforçant et en simplifiant les pouvoirs de sanction du maire.

créer une éco-contribution sur les produits non recyclables, à forcer à l'éco-conception des produits, à renforcer la lutte contre le gaspillage alimentaire ou encore à améliorer le futur traitement des biodéchets. En conclusion, je dirai que du chemin reste à parcourir,

Bien sûr, d'autres textes ont traité partiellement ces sujets, mais la notion d'économie circulaire est apparue relativement récemment. Cette notion recouvre en réalité une approche ou des pratiques basées uniquement sur le bon sens. Bien sûr, des citoyens, des collectivités, des entreprises, des associations, des parlementaires sont sensibles à ces thématiques, se sont investis par le passé et ont pris de nombreuses initiatives. Bien sûr, les attentes autour de ce texte sont fortes et légitimes. Il nous revient de traduire dans la loi de façon subtile et équilibrée cette aspiration collective. Ce projet de loi est issu d'une large concertation de plusieurs mois qui a regroupé de nombreux acteurs du secteur- entreprises, associations, collectivités ... -et qui a débouché sur la publication de la feuille de route pour l'économie circulaire. Avec Hervé Maurey, président de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, nous avons craint- nous l'avons écrit -que ce projet ne soit pas à la hauteur de cette concertation. Il ne semblait pas concevable qu'un projet aussi attendu ne soit composé que d'ordonnances et ne puisse pas faire l'objet d'un débat réel dans notre hémicycle. notre hémicycle. Nous sommes satisfaits de voir que nos remarques ont été entendues. Nous avons bel et bien un projet de loi qui nous a permis de débattre en commission et nous allons poursuivre nos échanges durant les prochains jours. À cet égard, je me dois de saluer le travail de la rapporteure, Marta de Cidrac, qui a permis, avec les contributions de nos collègues, de donner au texte une autre dimension. Et, contrairement à ce que vous avez déclaré dans, madame la secrétaire d'État, je pense que les sénateurs n'ont pas été frileux

Parmi les nombreux sujets abordés, il en est un qui concerne très directement les collectivités locales, c'est celui de la gestion et du traitement des déchets. J'ai la conviction, comme l'a démontré

J'ai pu l'éprouver dans l'intercommunalité que j'ai eu l'honneur de présider et au niveau d'un département comme celui de la Vendée, qui obtient des résultats très positifs en termes de tri et de performance. En incluant les collectivités qui ont engagé des études préliminaires, 16 millions de Français sont ou seront concernés par la tarification incitative- c'est insuffisant. Une incitation forte en faveur des collectivités optant pour ce système permettrait d'accélérer le développement de ce modèle vertueux- cette mesure avait d'ailleurs été suggérée dans les cinquante propositions de la feuille de route. Avec l'élargissement des consignes de tri, les performances s'améliorent. La question du plastique ne se cantonne pas aux seules bouteilles. Comment s'appelle le geste de tri qui consiste à mettre dans un sac jaune ou un point d'apport volontaire ses bouteilles ou produits plastiques, si ce n'est une consigne non marchande ? L'économie circulaire, c'est aussi la création de nouveaux gisements d'emplois. J'en veux pour preuve le développement du secteur du réemploi et de la réparation, qui compte désormais 6 700 structures en France et emploie 34 000 personnes, ce qui est considérable. Le volume de biens réemployés ou réutilisés est passé en trois ans de 780 000 tonnes à 1 million, soit une augmentation de plus de 28 %. Avec 100 millions de biens échangés en 2017 des plateformes internet ou des recycleries, les Français sont de plus en plus nombreux à opter pour des biens déjà utilisés. Une seconde vie, voire des vies multiples, s'offre à de nombreux objets et équipements.

De nombreuses entreprises ont investi dans l'économie circulaire avec l'idée que produire à partir de matières recyclées doit coûter moins cher que d'en extraire de nouvelles, ce qui paraît logique. De nombreuses barrières, comme le faible cours de certaines matières premières, ralentissent le développement du recyclage. Là encore, des dispositifs incitatifs devront être mis en place. Il reste à écrire de nouvelles pages au-delà de ce projet de loi. Toutefois, je suis convaincu que nos débats, sous la houlette de notre rapporteure et avec la bienveillance de Mme la secrétaire d'État et du Gouvernement, enrichiront ce texte d'une manière équilibrée et permettront à la France de devenir un modèle en matière d'économie circulaire.

à nous interroger sur la manière d'atteindre les objectifs de lutte contre la pollution de notre planète. Ainsi, alors que nous sommes tous d'accord pour reconnaître l'urgence d'un sursaut, nous sommes face à un texte qui prévoit des normes et des délais traduisant une méconnaissance de la vie des entreprises et des logiques économiques qui prévalent dans le monde. Prenons l'article 1 et ses obligations d'étiquetage ou de marquage des produits l'incorporation de matière recyclée, l'emploi de ressources renouvelables, la durabilité ou la réparabilité. Pour des exemples concrets, je vous invite à visiter la Cité de l'économie, qui vient d'ouvrir à Paris. L'un des ateliers montre, pour différents produits, le nombre incroyable de fournisseurs venant du monde entier pour des produits aussi simples, par exemple, qu'un pot de yaourt produit en France, dont la colle servant à sceller le couvercle en plastique peut provenir d'Asie. Pensez-vous que les producteurs français, notamment les plus modestes, vont être en mesure, d'ici à un an, d'obliger tous leurs fournisseurs à leur transmettre des informations aussi exhaustives, techniques et complexes à déterminer que celles requises par l'article 1 ? Fort heureusement, le texte adopté en commission prévoit un délai supplémentaire d'un an pour l'entrée en vigueur de cette mesure, comme pour celles des articles 2 à 4. Un autre facteur de découragement de nos entreprises vient de notre tendance à surtransposer les directives européennes. Comme l'a rappelé notre collègue Pierre Médevielle au nom de la commission des affaires européennes, les mesures de transposition partielle du projet de loi sont complétées par des obligations purement nationales, c'est-à-dire des obligations que le droit européen n'impose pas. C'est très bien d'être ambitieux en matière de protection de l'environnement, mais cela ne doit pas empêcher de prendre en compte les conséquences économiques de la surtransposition en matière de normes applicables aux entreprises françaises. C'est d'ailleurs ce que nous disons très souvent aussi pour l'agriculture. Avec la délégation aux entreprises, nous rencontrons en permanence des dirigeants qui nous expliquent que leurs concurrents européens, auxquels des normes moins contraignantes s'appliquent, ne cessent de gagner des parts de marché en France.

S'il y a un message que je souhaiterais faire passer- nous ne cessons de le rappeler avec mes collègues de la délégation aux entreprises -, c'est de légiférer en prenant en compte l'impact pour les entreprises, en particulier pour les TPE et les PME. Trop souvent, les projets de loi prévoient des mesures dont les modalités et les délais de mise en oeuvre sont totalement déconnectés de la réalité des processus de production. Pourtant, je voudrais rappeler que beaucoup de nos entreprises sont vertueuses. C'est le cas notamment du secteur du BTP, qui devrait atteindre l'objectif de 70 % du taux de valorisation de ses déchets. Nos artisans s'organisent déjà et les PME se mobilisent, mais tous nos chefs d'entreprise sont en permanence déstabilisés par des contraintes irréalistes qu'on leur impose de façon rigide. Enfin, certains d'entre vous ont pu voir les reportages du journaliste Hugo Clément qui montrent des déchets plastiques de produits français ayant suivi le cheminement du recyclage dans des décharges sauvages en Malaisie quel scandale, alors que nos entreprises ont déjà réalisé des efforts considérables pour mieux produire, alors que les citoyens ont adopté des comportements plus responsables et que les collectivités territoriales se sont mobilisées en faveur du tri sélectif Ces images montrent bien que l'on ne peut appréhender la question de l'économie circulaire sans prendre en compte et contrôler le devenir des déchets jusqu'au bout de la chaîne.

C'est bien la logique que nous devons avoir toujours en tête : une mesure qui paraît vertueuse peut en réalité entraîner des conséquences néfastes, indépendantes de notre volonté nationale de bien faire.

aujourd'hui, face à l'épuisement des énergies non renouvelables et des ressources naturelles, face au réchauffement climatique et à l'augmentation de la population mondiale, l'économie linéaire est incapable de répondre aux enjeux environnementaux et sociétaux du monde. Il nous faut, et c'est une urgence, accélérer cette vision circulaire que n'aurait pas reniée en son temps Lavoisier- avant de se faire couper la tête, comme d'autres ... -, quand il énonçait : « Rien ne se perd, tout se transforme ». C'est aujourd'hui d'une actualité saisissante. Notre défi consiste donc à participer activement à cette mutation et à repenser non seulement les méthodes de production, mais aussi la distribution et les comportements des consommateurs. Il faut que chacun prenne conscience du virage à prendre. En ce sens, nous ne pouvons que saluer ce projet de loi, qui vise à apporter des solutions durables et crédibles. Nous y souscrivons en partie, à condition qu'il soit suivi d'effet.

L'objectif à atteindre est bien de responsabiliser les metteurs sur marché dès l'amont, d'encourager les systèmes vertueux, de mieux informer le consommateur pour qu'il développe les bons gestes afin de concourir à une collecte de qualité, mais aussi d'améliorer le système de tri et de recyclage. Cependant, il était primordial, avant toute chose, de favoriser la notion de réemploi et de valorisation, car le texte, dans sa rédaction initiale, n'était centré, me semble-t-il, que sur la question de la gestion des déchets. Or le réemploi, défini comme toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus, est lui aussi essentiel à l'économie circulaire et peut engendrer une véritable économie sociale. Nous le voyons par exemple avec les meubles et les vêtements. Il est également nécessaire de réduire les déchets à la source et de privilégier l'éco-conception, car nous ne pouvons plus aujourd'hui nous permettre de décorréler l'analyse d'un produit de celle de son cycle de vie, qui comprend à la fois sa fin de vie, son utilisation et les différentes étapes nécessaires à sa production. À ce titre, la réforme et l'extension des filières à responsabilité élargie du producteur s'avèrent plus que jamais nécessaires. Je rappellerai que le Sénat a toujours été en pointe sur le sujet des REP.

et de concentrer nos efforts vers le hors foyer largement perfectible. Gageons que vous partagerez notre vision ! Il faut enfin une information lisible et claire pour le consommateur, et, bien évidemment, nous ne pouvons que souscrire aux simplifications proposées. Attention toutefois à ne pas déstabiliser nos entreprises qui interviennent sur le marché européen et qui seraient obligées de développer plusieurs emballages selon le marché, puisque, aujourd'hui, de nombreux pays européens continuent à rendre obligatoire le logo « point vert ». À cet égard, j'en appelle expressément au bon sens, qui voudrait que ce logo puisse continuer à être apposé sur l'emballage si celui-ci est multilingue. En conclusion, j'insisterai sur le fait que c'est bien de la mise en commun des synergies et des actions de toute la chaîne de valeur que dépend la réussite de ce passage à une économie de valorisation. Au fond, il s'agit ni plus ni moins d'un projet politique qu'il faut avoir le courage de porter. La discussion

dire à Mme la secrétaire d'État que j'ai été extrêmement surpris par ses propos, ce matin, dans la presse régionale et sur une radio de service public. Certains orateurs s'en sont

je fais le choix de ne pas vous répondre, parce que, vous le savez aussi bien que moi, vous m'avez à plusieurs reprises invectivée dans les médias.

des objectifs précis et chiffrés, afin d'instituer un circuit de consommation de nature à faire disparaître, à terme, l'empreinte de nos déchets. C'est pourquoi, aux prémices de l'examen de ce texte, il m'apparaît indispensable de prévoir dans la loi un objectif stratégique global et ambitieux de réduction de nos déchets ménagers assimilés et de nos déchets économiques hors secteur du bâtiment.

le présent amendement, tout en reconnaissant l'objectif de la politique nationale de prévention et de gestion des déchets ménagers mentionné dans le code de l'environnement, vise à lui adjoindre un objectif quantitatif sur le réemploi afin de concrétiser une telle démarche. Aujourd'hui, seules 940 000 tonnes de déchets ménagers sont réemployées sur 37,7 millions de tonnes, et 9,3 millions de tonnes de biens en fin de vie sont susceptibles de réemploi.

le recyclage- on prendra le verre comme exemple vraiment efficace -, la réutilisation ou valorisation- on pense au compost -ou le réemploi. Parmi ces trois piliers, le réemploi est, de loin, celui qui répond le mieux à un objectif d'économie circulaire ne pas produire de déchets. En donnant une seconde vie aux objets, on ne ponctionne ni ressources supplémentaires ni énergie dans une industrie de transformation, et on n'émet pas de gaz à effet de serre. Mieux encore, le réemploi est une activité profondément sociale. Que l'on parle de dons, de vente à très bas coût de produits de seconde, voire de troisième main, d'aide à la réparation pour éviter d'acheter neuf, le réemploi est un mode de consommation sobre et abordable pour toutes et tous. Encore mieux, le réemploi permet l'emploi. Les acteurs du réemploi- associations et entreprises de l'économie sociale et solidaire -créent plus d'emplois que n'importe quel autre mode de gestion des déchets. On estime ainsi que là où l'incinération de 10 000 tonnes de déchets crée trois emplois, le réemploi de 10 000 tonnes de « déchets » en crée, lui, 800. Dans notre société au chômage structurel, c'est une piste à étudier Avec cet amendement, nous proposons ce qui nous semble le minimum que l'on puisse attendre d'un projet de loi s'intitulant « lutte contre le gaspillage et économie circulaire », à savoir l'instauration d'un objectif national de réemploi de nos déchets. Qui plus est, nous proposons un objectif particulièrement modeste, à une échéance presque lointaine, à savoir 5 % du tonnage de nos déchets à horizon de 2030. Cela revient tout de même à doubler l'existant ; c'est dire si nous avons des progrès à faire. La

Sur les 37,7 millions de tonnes de déchets ménagers que la France produit annuellement, seuls 2,5 % sont réemployés ou réutilisés. Des marges de manoeuvre existent donc en la matière, puisque le réemploi et la réutilisation, au sommet de la hiérarchie des modes de traitement des déchets, permettent de prolonger la durée de vie des produits, d'économiser nos ressources et de participer à la réduction des déchets. L'objet du présent amendement est donc de doubler le pourcentage des déchets ménagers réemployés ou réutilisés en 2030.

C'est très difficile de mesurer la part de déchets qui font l'objet d'une simple réparation, la part de déchets qui viendraient de produits achetés sur une plateforme en ligne ou la part

même si, dans l'esprit, je pense que vous avez absolument raison de vouloir souligner l'importance du réemploi et de la réutilisation.

il me paraît important d'inscrire notre action dans le cadre d'orientations claires, précises et chiffrées. L'impact de l'usage du plastique sur nos écosystèmes n'est plus à prouver. Aussi, nous souhaitons limiter la circulation d'emballages en plastique à usage unique sur le marché français. Pour ce faire, nous proposons d'inscrire dans la loi deux objectifs stratégiques : réduire la présence de ces plastiques de 50 % entre 2020 et 2030, et les 50 % restants entre 2030 et 2040. Quel

contre la pollution plastique. Nous avons d'ailleurs déjà commencé à engager toute une série d'actions très concrètes en ce sens. Je pense, par exemple, au pacte national sur les emballages plastiques, qui a réuni des industriels et des acteurs de la grande distribution, lesquels devront rendre des comptes chaque année. Le but est d'avoir 100 % d'emballages recyclés d'ici à 2025 et de lutter contre la prolifération de plastique et le suremballage dans les années à venir, avec des ONG qui vérifient chaque année où nous en sommes. Le Premier ministre

en matière de réduction de nos déchets, particulièrement ceux en plastique. Il s'agit, madame la secrétaire d'État, de donner un véritable cap à votre projet de loi, qui, avant son passage au Sénat, ne fixait finalement aucun objectif clair en matière de réduction de notre consommation de plastique. La France est pourtant le premier producteur européen de déchets plastiques, avec 4,5 millions de tonnes produites chaque année. À ce titre, nous avons une responsabilité forte et nous devons avoir une véritable ambition en matière de lutte contre cette pollution. à l'heure des bouleversements climatiques que nous connaissons et de la disparition des espèces animales comme végétales, il est temps de changer de modèle de société et d'engager une véritable mutation dans notre façon de consommer, mais aussi de produire. Par cet amendement, nous ne proposons pas de fixer tel ou tel taux à atteindre dans cinq ou dix ans, ce qui aurait suscité des débats, des divergences, voire des oppositions. Nous proposons de poser un cadre juridique et politique pour se donner les moyens d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés à l'article L. 541-1 du code de l'environnement, notamment à l'occasion de la loi de transition énergétique de 2015. Il sera nécessaire que ces objectifs intègrent une dimension économique et sociale en accompagnant les entreprises dont la reconversion serait inévitable. Il n'est pas question de laisser des milliers de salariés sur le bord de la route, mais au contraire d'engager collectivement une véritable révolution de notre modèle de production et de consommation vers un système sobre, plus vertueux et respectueux de l'environnement. C'est l'objet du présent amendement.

Les pouvoirs publics doivent mettre en oeuvre un plan ambitieux de lutte contre la pollution des plastiques dans l'environnement. C'est tout à fait en accord avec les objectifs que nous venons de nous fixer. L'avis de la commission est donc favorable.

Ces équipements se développent lentement, mais ils ont déjà un impact significatif sur la gestion des déchets, avec plus de 160 000 tonnes de déchets réemployés ou recyclés, soit plus de 500 tonnes annuelles par équipement. Je ne reprendrai pas tout l'argumentaire que j'ai développé à mon amendement précédent, mais j'indique que cette activité, en plus d'être particulièrement vertueuse d'un point de vue écologique, est créatrice d'emploi, de lien social, est un vecteur d'éducation populaire et de dynamisme local. Chaque élu local ayant vu naître une ressourcerie sur son territoire peut mesurer l'ensemble des bénéfices qu'elle apporte aux communautés locales. Seulement, pour avoir un impact national, le réseau d'équipements de réemploi doit fortement se densifier. En cohérence avec la compétence déchets, nous proposons de mettre en place au moins un équipement de réemploi par EPCI et, pour faire face aux volumes qui peuvent rapidement devenir importants, au moins un par tranche de 22 000 habitants en zone urbaine. Ces 2 500 ou 3 000 nouveaux équipements permettraient d'employer des dizaines de milliers de personnes et de réutiliser et de favoriser des centaines de milliers de tonnes de déchets. Cela permettrait notamment de réduire la pression sur les déchetteries, dont le maillage est de 1 pour 14 000 habitants. Quel

Toutefois, la planification que vous proposez pour le déploiement d'un grand nombre de ressourceries et de recycleries dans chaque EPCI et par tranche de 22 000 habitants sans étude d'impact ni évaluation préalable me paraît délicate à inscrire dans la loi et pourrait conduire à un surdimensionnement. C'est la raison pour laquelle l'avis est défavorable. Quel est l'avis du Gouvernement

qui repense nos modes de production et de consommation afin de préserver nos ressources et de limiter la production des déchets. À ce titre, les emballages revêtent une symbolique très importante, car ils sont une source de pollution majeure et sont présents en permanence dans notre quotidien. Nous proposons ainsi d'atteindre un objectif de 85 % d'emballages recyclables sur le marché avant 2025, laissant ainsi cinq ans aux industriels pour trouver des substitutions aux emballages les plus difficiles à recycler. Au total, nous nous fixons donc un objectif de dix ans pour y parvenir totalement, des délais qui semblent largement suffisants aux industriels pour s'adapter et envisager des modèles de substitution. Comme vous le constaterez, nous visons tous les emballages et non pas seulement ceux qui sont en plastique, même si nous savons que 45 % de la consommation de plastiques en France concerne les emballages. C'est pourquoi notre amendement n'est pas redondant avec l'article 1 1 A introduit en commission. Bien évidemment, l'objectif que nous vous proposons n'est qu'une étape, car un emballage recyclable n'est pas nécessairement recyclé. C'est par exemple le cas des emballages en plastique : si 50 % de ceux qui sont mis sur le marché sont recyclables, seuls 26 % sont recyclés.

par l'objectif de 100 % de plastiques recyclés à horizon de 2025 et par l'objectif de réduction de mise sur le marché d'emballages plastiques à usage unique. En outre, ces objectifs de recyclabilité pourront être inscrits dans le cahier des charges de l'éco-organisme compétent sur cette filière,

est à M. Roland Courteau, sur l'article. Les plastiques sont partout : dans l'air, dans l'eau, dans les aliments, dans nos organismes, sur nos tables. On trouve jusqu'à 100 000, voire 900 000 microplastiques par kilomètre carré dans certaines zones de la Méditerranée. On en trouve dans les Pyrénées jusqu'à 1 500 mètres d'altitude. De nouvelles pollutions émergent, dont celle des microfibres provenant de nos vêtements, des microbilles, issus des produits de gommage cosmétique. Il s'agit là de véritables bombes à retardement, dont j'avais fait état d'ailleurs dans un rapport de l'Opecst, qui ciblait les pollutions en Méditerranée. Sur ce bassin méditerranéen, la France est le plus important producteur de déchets plastiques : 80 000 tonnes sont rejetées dans la nature et 11 000 finissent en Méditerranée. Notez que la France a produit, jusqu'en 2016, 18 milliards de sacs en plastique ! À l'instant, je parlais de bombe à retardement. Et pour cause En mer, notamment, les macrodéchets se fragmentent en microdéchets, puis en nanodéchets qui sont absorbés par les espèces constituant le début de la chaîne alimentaire. Dans certaines zones de la Méditerranée, il y a autant de microplastiques que de planctons Question : jusqu'où ces contaminations peuvent-elles s'infiltrer dans la chaîne alimentaire ? Selon une étude, l'être humain avalerait 5 grammes de plastique par semaine, soit l'équivalent d'une carte de crédit. Le coût des dommages environnementaux est chiffré. Quant à la perte pour l'économie bleue française, elle s'élèverait aux environs de 73 millions d'euros. Et que dire du coût sanitaire ? Que deviennent en effet dans notre organisme les substances telles que les phtalates, le bisphénol, substances mutagènes, reprotoxiques ? C'est une bonne question. Dès lors, 100 % de recyclage à l'horizon de 2025, comme le prévoit cet article, me paraît hautement nécessaire, et je salue cette initiative. C'est bien, mais il faut aller plus loin encore. Le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas. Il nous faut donc aussi concentrer les efforts sur la réduction à la source des plastiques et sur la prévention et la remise en cause de nos modes de consommation. C'est le sens d'ailleurs des amendements que nous venons d'adopter. Deux questions, madame la secrétaire le G7 de Biarritz devait bâtir une coalition pour lutter contre ces pollutions. Qu'en est-il ? Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus ? Et qu'a-t-il été décidé à Marseille sur ce point par l'Union internationale pour la conservation de la nature

1 A est supprimé. J'informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion sur le projet de loi relatif à la modernisation de la distribution de la presse est parvenue à l'adoption d'un texte commun.